et le vote par scrutin public sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

le patron du Programme alimentaire mondial (PAM) a, cette semaine, alerté sur la très grave sécheresse qui frappe actuellement Madagascar, entraînant la première famine sur le continent africain depuis longtemps, sans qu'aucune guerre ou conflit n'en soit à l'origine. Cette situation n'est liée qu'à plusieurs années de sécheresse consécutives, ce qui fait dire à la directrice de la branche locale du PAM qu'il s'agit de la première famine totalement due au réchauffement climatique.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous y voilà

est devant nous, mes chers collègues, et nous devons y faire face avant qu'il ne soit trop tard. Si nous voulons être capables de réussir, de vivre et de nous développer, nous devons ne plus attendre et ne plus nous payer de mots. Il faut agir, agir et encore agir alors que nous débattions de ce projet de loi, le sixième rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a fuité dans la presse. Les experts s'y alarment des impacts dévastateurs que le réchauffement aura sur notre planète dès les prochaines décennies. Ils rappellent l'urgence d'une action politique ambitieuse et résolue en faveur du climat, face aux conséquences irréversibles d'une attitude attentiste. Le rapport apporte aussi une note d'espoir. Il affirme que l'humanité peut encore changer le cours des choses, à condition d'opérer une « transformation radicale des processus et des comportements à tous les niveaux Mais nous savons tous, et nos débats sont là pour en attester, que cette radicalité ne peut être obtenue sans l'adhésion massive de nos concitoyens, au risque d'échouer lamentablement et de se retrouver dans le mur. Méfions-nous de celles et ceux qui appellent au grand dérangement, comme d'autres avant eux à de grands bonds en avant ; ils mènent à l'autoritarisme et à la misère collective. collective. Soyons donc clairs, nets et précis. Admettons que la France prend toute sa part dans la démarche, y compris en étant moteur des autres parties prenantes. Depuis 2017, elle mène une action résolue, concrète et ambitieuse, qui lui permet de s'affirmer comme un leader de la lutte contre le réchauffement climatique dans le monde.

l'inscription dans la loi de la neutralité carbone d'ici à 2050 ; la mise en place d'un plan Biodiversité doté de 600 millions d'euros et portant 90 mesures, parmi lesquelles figure l'interdiction de la plupart des produits plastiques à usage unique ; l'arrêt du projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la fermeture de la centrale de Fessenheim et l'abandon du projet Montagne d'or en Guyane.

Nous ne croyons pas à une écologie qui viendrait simplement d'en haut. C'est ce qui a inspiré la création de la Convention citoyenne pour le climat, dont l'essentiel des propositions est traduit dans ce projet de loi. Avec ce texte, l'ambition affichée est de mettre un terme à un ensemble de pratiques incompatibles avec nos ambitions climatiques la fin de l'étalement urbain sans limite, l'interdiction de la mise en location des passoires thermiques, l'interdiction des vols domestiques pour lesquels il existe une alternative moins émettrice en CO2 pour un temps de trajet inférieur à 2 heures 30, la régulation de la circulation des voitures les plus polluantes dans nos grandes villes. Mais ne nous y trompons pas, l'ampleur du défi, rappelée par le GIEC, rend toute solution nationale largement insuffisante. La réponse ne pourra être qu'européenne et internationale. La France, à nouveau, prend toute sa part. Elle montre l'exemple et entraîne ses partenaires européens, en promouvant une action internationale dans nos relations bilatérales comme multilatérales. Ce texte, je le disais en ouverture de mon propos, a fait l'objet d'un examen minutieux et approfondi dans nos commissions respectives et en séance. Le mérite premier en revient aux présidents de commission et aux rapporteurs, qui ont réalisé un travail remarquable et remarqué, dans un souci réel d'écoute, même si nous ne partageons pas toutes leurs conclusions et propositions. Mais c'est aussi la force de la démocratie que de pouvoir confronter, dans un climat apaisé, points de vue et propositions. Oui, nous ne partageons pas toutes les options retenues par le Sénat, considérant qu'elles ne sont pas les plus à même de répondre aux enjeux qui sont face à nous. Nous pourrions ainsi évoquer le refus du Sénat de basculer vers le dispositif du « Oui pub », les ambiguïtés manifestes de la majorité sénatoriale dès lors que l'on parle d'énergies renouvelables décarbonées, le manque de volonté patent pour mettre en place les zones à faibles émissions (ZFE), la baisse de TVA à 5,5 % pour les transports collectifs de voyageurs

Nombre de collègues, à droite et à gauche de notre hémicycle, ont regretté le manque d'ambition du texte. Bien au contraire, ce projet de loi se fonde sur la confiance envers nos concitoyens et sur la responsabilisation des acteurs de la société. Ces éléments sont les préalables de l'appropriation des enjeux écologiques par l'ensemble de la société. Avec ce texte, nous faisons le pari du bon sens des Français. Une série de dispositifs les concerne, en tant que consommateurs, usagers de la route, propriétaires de logement, clients de la restauration collective, dirigeants d'entreprises.

La volonté politique portée par ce texte est très clairement exprimée. Elle concilie écologie, préoccupations sociales et économie de manière pragmatique, afin de répondre aux défis cruciaux de notre temps. Députés et sénateurs connaissent désormais le chemin à suivre pour atteindre les objectifs que nous savons communs. Et parce que nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais que nous reconnaissons la qualité du travail accompli et certaines ouvertures qui ont pu être faites, le groupe RDPI s'abstiendra sur le texte. La parole

nos niveaux actuels d'adaptation seront insuffisants pour contrer les menaces- événements extrêmes, stress hydrique, maladies, déclin des cultures de base et de la valeur nutritionnelle des aliments également que l'humanité ne pourra se remettre d'un changement climatique majeur, même si ce constat n'est pas inéluctable. Il est encore possible de transformer radicalement les comportements à tous les niveaux : individus, communautés, entreprises, institutions et gouvernements. Mais avons-nous le même niveau de lecture de ces données ? Faisons-nous confiance à nos experts ? Nous avons, depuis des mois, reçu de très nombreuses sollicitations sur ce projet de loi. L'adhésion n'est pas là. Les résistances sont fortes. Pourtant, une part croissante de nos concitoyens prend toute la mesure de l'ampleur du défi. J'entends et je souscris aux arguments selon lesquels la France ne peut, à elle seule, assumer la charge de la lutte contre le changement climatique et se placer systématiquement en situation de subir la concurrence déloyale, car de l'économie dépend également notre survie. Je le dis souvent dans cet hémicycle, l'échelle européenne doit être pleinement mobilisée et privilégiée. Mais la France doit prendre ses responsabilités. C'était le sens des amendements symboliques qui ont été votés en préambule de nos débats. Notre rôle premier, en tant qu'élus, est de sensibiliser, de convaincre et d'accompagner pour déclencher l'acceptation sociale. La loi ne peut pas tout et tel n'est pas son rôle. Le taux d'abstention lors des élections départementales et régionales démontre que l'adhésion à nos projets politiques n'est pas acquise. Les démarches vertueuses doivent être encouragées. Les dispositions du projet de loi relatives à l'amélioration de l'information du consommateur sont bienvenues. L'existence de pratiques commerciales trompeuses en matière environnementale prouve que l'intérêt des citoyens se tourne davantage vers les biens et services les plus respectueux de l'environnement.

L'accompagnement des ménages modestes, mais aussi des classes moyennes, en matière de transports est également primordial dans un contexte d'extension des restrictions à la circulation. Le Sénat a fait oeuvre utile par la mise en place d'un prêt à taux zéro pour l'acquisition de véhicules et de poids lourds peu polluants, l'établissement d'un taux de TVA à 5,5 % pour les billets de train ou encore l'instauration d'un dispositif de fixation d'un prix plancher pour certains billets d'avion. Le titre relatif au logement constitue notre plus grande déception. La massification de la rénovation énergétique des bâtiments est compromise. Les dates retenues pour qualifier d'indécentes les passoires énergétiques

si elle représente un quart de nos émissions de gaz à effet de serre, elle constitue également un point central en raison du processus de captation de dioxyde de carbone par le sol. Il ne peut y avoir de lutte contre le réchauffement climatique sans les agriculteurs. Je tiens ainsi à saluer toutes les mesures destinées à valoriser les produits locaux, durables et de qualité, renforcées par le Sénat. Mais l'urgence est avant tout de récompenser les bonnes pratiques et d'assurer le partage de la valeur, c'est-à-dire un revenu correct pour À défaut, les investissements de ces derniers pour l'agroécologie risquent de les pénaliser. Je me réjouis de l'adoption de l'amendement de Franck Montaugé, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, inscrivant dans la loi la reconnaissance et la valorisation des externalités positives de l'agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d'aménagement du territoire. Dans un texte comprenant un titre entier dédié à l'artificialisation des sols, je regrette que la protection des terres agricoles n'ait pas été approfondie. J'avais déposé un amendement, déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution, visant à sacraliser la vocation agricole des terres qui ont bénéficié, à ce titre, d'aides publiques locales, nationales, voire européennes.

Vous cautionnez donc collectivement, mes chers collègues, que des terres agricoles irriguées, par exemple, grâce à des financements publics, soient urbanisées. Je ne comprends pas cette contradiction : tout le monde est d'accord pour défendre l'agriculture, mais personne ne veut graver dans le marbre la protection durable des terres agricoles. En ce qui concerne le droit pénal de l'environnement, le Gouvernement est passé à côté de la réforme d'ampleur qui aurait dû aboutir à sa simplification et, ainsi, à sa pleine effectivité. Le choix a été d'opérer par petites touches de complexité supplémentaire sans créer, comme le recommandaient de nombreux juristes, un véritable délit de mise en danger de l'environnement et un délit générique visant à sanctionner l'ensemble des atteintes à l'environnement. Le caractère durable de ces atteintes, exigé par les articles 67 et 68 du projet de loi, rend ces délits inapplicables. Quant à la reconnaissance de l'écocide au niveau international, nous serons vigilants. Si nos idéaux se confrontent aux réalités d'une économie mondialisée, ne laissons pas cette dernière les briser définitivement. La solution est sans nul doute dans la concertation et le compromis démocratique. Malgré les critiques acerbes qui ont été exprimées ici et là, l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat doit être étudiée et perfectionnée. Cela n'enlèvera rien à la légitimité de la démocratie représentative ; bien au contraire, cela la confortera dans ce qu'elle a de plus noble : la représentation de l'intérêt général. Certes, c'est une méthode complexe. Mais il est primordial de la développer. Car,, c'est l'acceptabilité qui est visée. Je regrette que les limites de l'exercice n'aient pas été fixées dès le départ. Il était illusoire de faire croire aux participants que toutes les préconisations seraient suivies en l'état. C'est nier le débat parlementaire, essentiel dans le processus, et c'est susciter des frustrations. Pour conclure, après ces deux semaines de débats, il me vient surtout à l'esprit un dessin de Xavier Gorce de 2017. On y voit l'un des pingouins affirmer : « C'était mieux avant. » Lorsque l'autre lui demande : « Quand ? », il répond : « Quand je croyais que ce serait mieux après. » Mes chers collègues, pour que le monde soit mieux après, les efforts doivent être engagés dès maintenant. Ce texte manque d'audace et d'ambition, raison pour laquelle je m'abstiendrai, comme la majorité de mon groupe.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il est déjà minuit pour notre planète, pour l'humain, pour le vivant. Le vieux monde est en train de s'écrouler, la planète se dégrade chaque jour de façon irrémédiable, les espèces disparaissent par centaines chaque année, des populations entières voient leur habitat en danger, voire dévasté, et malgré cela nous regardons ailleurs. Les catastrophes climatiques ne sont plus des phénomènes isolés et lointains. Elles nous touchent plus vite, plus fort et plus souvent, mais nous continuons de regarder ailleurs. Selon les experts du GIEC, lorsque les enfants nés cette année auront 30 ans, le monde sera déjà irrémédiablement dégradé, soumis aux pénuries d'eau, aux exodes, à la malnutrition et à l'extinction des espèces. En 2050, que diront nos enfants et petits-enfants de nous ? Que diront-ils de notre inaction climatique, alors que nous savions et que nous n'avons rien fait ou si peu ? Nous refusons d'accepter le changement vital qui s'impose à nous, changement de mode de pensée, de mode de vie et, surtout, de ce système capitaliste qui épuise l'humain, le vivant, les ressources et la planète au profit de quelques-uns et au détriment du plus grand nombre. À la place, on nous dit que le chemin est long, qu'il faut maintenir nos efforts. Ces derniers ressemblent à de petits sparadraps avec lesquels on tenterait d'arrêter une hémorragie massive. Nous sommes pourtant la dernière génération de femmes et hommes politiques à pouvoir agir avant qu'il ne soit trop tard pour les limites planétaires,

vous n'avez voulu écouter que vous-mêmes et vos peurs d'une rupture radicale, pourtant nécessaire. Vous ignorez celles et ceux qui se mobilisent : les associations, les syndicats, la jeunesse, jusqu'aux membres de la Convention citoyenne pour le climat que vous aviez missionnés. Les propositions qu'ils ont construites, y mettant du temps, de la réflexion, de l'énergie, mais aussi de l'espoir, vous les piétinez avec ce texte ! Le mot d'ordre des débats sur ce projet de loi fut l'évitement.

La suppression des aides au maintien en agriculture biologique ne sera pas compensée et les aides au développement des protéines végétales ne seront pas suffisantes pour mettre fin aux importations de soja, destinées à l'alimentation des élevages industriels. Avec le goulag, c'était mieux ! Que dire, enfin, de l'attentisme interminable face au fléau des engrais azotés ? Nous avons discuté des heures sur les repas bio ou végétariens, alors que se multiplient les accords de libre-échange mortifères, responsables de l'augmentation du trafic de marchandises, de la déforestation, du dumping social et écologique. Vous les maintenez sans sourciller et évitez, une fois encore, de vous confronter à cette question. Ensuite, vous avez évité de prendre en compte les engagements internationaux de la France en fixant un objectif de diminution de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030,

% d'ici à 2030. Toutefois, selon le Haut Conseil pour le climat, ce texte n'engage aucun changement structurel nécessaire. En outre, une proportion élevée de ses dispositions voit sa portée réduite par un périmètre d'application limité. Le constat est sans appel : en l'état des mesures prises, la France n'atteindra pas ses objectifs. De la même manière, nous nous sommes émus des problématiques de partage des usages de l'eau, car nous savons que le stress hydrique est une donnée incontournable. Dans le même temps, le Gouvernement a accepté, voire orchestré, la privatisation de l'eau potable en France avec l'affaire Suez-Véolia. En ce qui concerne les entreprises et les banques, le Gouvernement et la majorité sénatoriale restent dans le déni. Pourtant, un rapport conjoint des Amis de la Terre France et d'Oxfam souligne l'absence d'engagement des établissements bancaires dans la transition énergétique. Pire, ces derniers soutiennent à hauteur de 100 milliards de dollars les entreprises actives dans les énergies fossiles. Il n'y a rien dans ce texte qui les contraigne à tendre vers la décarbonation de leurs activités. Enfin, et surtout, vous avez évité un élément fondamental : la justice sociale. Alors que les inégalités explosent, vous ignorez toujours les plus précaires, ceux qui seront les plus touchés par les crises à venir. Tout le monde attend que nous mêlions justice climatique et justice sociale. Nos concitoyens se soucient de l'état de la planète et aimeraient pouvoir la préserver. La transition doit donc être accessible à toutes et à tous. L'évitement a été total, du début à la fin, la commission déclarant même nos amendements irrecevables.

plus sur le service public ferroviaire et les trains d'équilibre du territoire (TET). Et la liste est encore longue ... Il faut reconnaître que le Sénat, sur certains points, a amélioré le texte initial initial : publicité pour les véhicules polluants, intégration des impacts sociaux et du respect des droits humains dans l'affichage environnemental, réduction de la TVA sur les billets de train à 5,5 % et exclusion d'entreprises qui ne satisfont pas à l'obligation d'établir un plan de vigilance de certains marchés. Toutefois, certains reculs sont inacceptables, comme en matière de zones à faibles émissions, alors que les morts prématurées liées à la pollution de l'air ne sont plus contestables. Et que dire de la gestion des installations de fret qui pourront être externalisées, actant un peu plus la casse de SNCF Réseau ? Il n'est plus possible de croire que, sans remise en cause du dogme de la concurrence libre et non faussée, ainsi que de l'idée d'un monde sans limites, nous puissions répondre aux enjeux climatiques et environnementaux. Oui, un texte qui porte l'ambition d'un changement de société doit mettre au coeur du débat les biens communs et le service public.

remercier les membres de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable pour leur engagement, en particulier ses rapporteurs, qui n'ont pas ménagé leurs efforts ces derniers mois. Je remercie également les rapporteurs des commissions saisies pour avis pour le travail collectif et complémentaire réalisé en bonne intelligence.

si la Convention citoyenne a démontré que certaines formes de démocratie directe ou participative pouvaient trouver une place dans la V République, elle n'a jamais eu vocation à se substituer au pouvoir législatif. Le Parlement a ainsi démontré qu'il n'abandonnerait pas son pouvoir de proposition et son droit d'amendement. Le texte qui nous arrivait de l'Assemblée nationale nous semblait manquer d'ambition et de pragmatisme. Nous doutions même de son effet climatique, tant il passait à côté de nos engagements européens rehaussés en décembre dernier. Nous regrettions aussi que ce projet de loi soit paradoxalement bavard sur des points de détail et muet sur des secteurs essentiels pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

d'ici à 2030, notamment parce qu'elles n'abordent pas les questions centrales que sont le mix électrique et la tarification du carbone. » Il est donc logique que le présent projet de loi reflète ces faiblesses originelles. Nous pourrons dès lors nous pencher autant que nous le souhaitons sur la question des échantillons commerciaux, des avions publicitaires ou demander pléthore de rapports. Pour ma part, qu'il est temps d'agir sur les principaux leviers qui nous permettront de rehausser l'effet climatique du projet de loi et, plus généralement, d'engager notre pays sur la voie de la neutralité carbone. Dans cette optique, je tiens à saluer les nombreux apports du Sénat, qui s'articulent autour de trois ambitions. Premièrement, supprimer les angles morts du texte. Je salue l'inscription dans le projet de loi de l'objectif de doublement des parts modales du fret ferroviaire et fluvial et la concrétisation de cette ambition la diminution de la TVA à 5,5 % sur les billets de train. Je salue également l'impulsion bienvenue pour nos forêts : il nous fallait optimiser leur rôle de puits de carbone, sachant qu'elles absorbent chaque année en France plus de 11 % de nos émissions de gaz à effet de serre. Deuxièmement, concilier économie, écologie et justice sociale. Je pense à la logique selon laquelle les aides à la rénovation énergétique doivent être davantage attribuées en fonction des revenus et non uniquement de la performance de la rénovation et au rétablissement du taux de TVA à 5,5 % sur les travaux de rénovation énergétique dans le logement social.

en créant des emplois non délocalisables, en réduisant les émissions polluantes et en améliorant la santé des populations. Troisièmement, défendre une écologie territoriale et pragmatique.

et dynamisé la politique alimentaire territoriale. Mes chers collègues, le Sénat a démontré son ambition écologique. Il n'est pas une assemblée ringarde qui passe à côté des grands défis de son temps.

« Ce que Paris conseille, l'Europe le médite ; ce que Paris commence, l'Europe le continue », disait Victor Hugo. En amont de la COP26 et de la présidence française de l'Union européenne, notre pays peut donner une impulsion climatique ambitieuse à ses partenaires européens- impulsion qui se retrouverait demain dans les accords commerciaux, par exemple en ce qui concerne la tarification carbone. C'est tout l'enjeu de cet amendement qui tend à réaffirmer les engagements climatiques européens et internationaux de la France, déposé par la plupart des groupes politiques du Sénat, à commencer par le groupe Union Centriste. Plus globalement, le groupe UC a pris toute sa part dans ce débat. Nous nous réjouissons d'avoir fait adopter en séance des amendements d'importance. Nous avons ainsi fait entrer dans le code minier la notion de « gestion minière durable acté la création d'un schéma directeur des itinéraires cyclables, inscrit le principe d'une modulation de l'écotaxe pour les poids lourds à faibles émissions ou encore fait adopter un principe de dérogation aux règles de la commande publique pour développer la rénovation énergétique des bâtiments publics. Fort de ces apports concrets, le groupe Union Centriste votera en faveur de ce projet

arc-boutée sur un savant discours construit autour de l'« écologie punitive »- belle trouvaille rhétorique pour justifier l'immobilisme. Pourtant, mes chers collègues, le contexte dans lequel se sont déroulés nos débats aurait dû nous convaincre de la responsabilité écologique qui nous incombe la canicule à Paris, les dérèglements climatiques récurrents, les fuites du nouveau rapport du GIEC anticipant des « retombées climatiques cataclysmiques » ou encore le rapport Tirole-Blanchard qui souligne la « menace existentielle » que fait peser le réchauffement Les signes annonciateurs sont là et nous continuons de disserter sur l'autorégulation des agents économiques, de multiplier les expérimentations sans définir de trajectoires claires, de ne pas entendre ce que nous disent les citoyens formés par les meilleurs experts que compte notre pays. À force de surplace, de communication, d'aveuglement devant les conséquences réelles du changement climatique, devant ce temps que nous laissons filer, nous construisons des usines à gaz et organisons notre propre impuissance, comme avec le démantèlement d'EDF, par exemple, au lieu de nous attaquer vraiment à la réduction des gaz à effet de serre. Comment voulons-nous revivifier notre démocratie si nous nous condamnons à l'inaction ? Lorsque le Gouvernement abaisse la stratégie nationale bas-carbone (SNBC), nous n'assumons pas notre leadership écologique, apparu au précédent quinquennat avec l'accord de Paris. Et pourtant, le ferment du nouvel universalisme français du XXI siècle consiste bien à lier l'écologie à la justice sociale. Le GIEC nous y invite : « Nous avons besoin d'une transformation radicale des processus et des comportements à tous les niveaux individus, communautés, entreprises, institutions et Gouvernement [ ...] Nous devons redéfinir notre mode de vie et de consommation ». Ce projet de loi y participe-t-il ? Malheureusement non, ou trop fébrilement. il ne s'agit d'être non pas alarmistes, mais réalistes. Nous ne pouvons que regretter que le Sénat, dans sa majorité, n'ait pas encore terminé sa mue écologique. Trop de vieux réflexes, trop de certitudes nous confinent encore à l'insécurité écologique. Si bien que toute une jeunesse, touchée par la faiblesse générale de nos débats, appelle aujourd'hui à ce que l'ensemble de la classe politique soit formée aux enjeux climatiques, tout comme le furent les 150 citoyens tirés au sort.

Nous pouvons tout de même nous réjouir de l'adoption de quelques-unes des propositions que nous semons depuis bientôt cinq ans- la patience a du bon. Je pense à l'introduction de critères sociaux dans l'affichage environnemental, au renforcement du contrôle des engagements des publicitaires

territoires ruraux. Il s'agit d'une avancée très importante, au même titre que l'introduction dans notre politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation de la nécessité de préserver nos agriculteurs de la concurrence déloyale des produits importés ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne.

Sans évaluation des impacts sociaux des mesures prises en termes de pouvoir d'achat et d'emplois, la transition écologique est condamnée à échouer, faute d'acceptabilité sociale.

Nier la dimension solidaire de la transition écologique ne fera que renforcer les inégalités face au réchauffement climatique. Je terminerai par une illustration très concrète de nos débats, qui démontre nos difficultés, en tant que groupe de l'opposition, à faire valoir le réalisme écologique

ne touchons surtout pas aux ultraprivilégiés ! -alors qu'il s'agit de défendre l'intérêt général et nos enfants ; ... Quelle caricature ! ... de l'autre, la droite de cet hémicycle, tout en repoussant l'interdiction de location des logements classés F,

Voilà l'écueil politique, les paradoxes de la communication et l'inertie auxquels nous sommes confrontés au moment d'enclencher la transition écologique et solidaire. Si le projet de loi contient des petits pas, il constitue un terrible aveu d'impuissance climatique et un véritable échec pour le Gouvernement. Alors que la Convention citoyenne pour le climat fut une très belle réussite démocratique, nous ne pouvons que regretter la faiblesse de sa traduction législative. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre le texte qui nous est proposé. La parole

Face aux intérêts court-termistes de quelques-uns, il nous invite à voir la transmission dans le temps long et à protéger ce qui fait notre bien commun. Si l'écologie nous concerne tous, la vague notion de climat et résilience en titre de ce projet de loi annonçait déjà un contenu conforme à un prêt-à-penser bien éloigné d'une clairvoyance écologique nouvelle. Confondre écologie et climat, c'est déjà laisser libre cours à l'idéologie qui fait de la taxation l'alpha et l'oméga d'un écologisme aussi punitif qu'inefficace. Ce projet de loi reflète le « en même temps » progressiste, friand de contradictions. Ce texte se contente de mesures néfastes ou de surface. Je pense en particulier aux éoliennes, véritable totem sacré de l'écolo-boboïsme : elles polluent nos sols avec des milliers de mètres cubes de béton, tuent nos oiseaux et font fuir la faune ; elles ont un bilan carbone déplorable, ruinent des milieux de vie, vie, défigurent les contours poétiques de nos paysages. Dans les Bouches-du-Rhône, le projet d'implantation de ces horreurs au pied de la merveilleuse montagne Sainte-Victoire, si chère à Cézanne et à tous les amoureux de ce que la nature nous a offert de plus beau, est un véritable crime ! Avec les parcs éoliens et solaires terrestres ou offshore, vous industrialisez et défigurez nos paysages, vous généralisez le retour aux centrales à gaz et à charbon pour un bilan écologique négatif. Il est donc important d'autoriser les maires à refuser l'implantation d'éoliennes sur leur commune. C'est ce qu'a fait le Sénat, dans sa grande sagesse- nous ne pouvons que nous en réjouir. Notre assemblée a aussi supprimé la notion de crime d'écocide, laquelle aurait pu se retourner contre votre chantier de forage d'éoliennes offshore en baie de Saint-Brieuc, madame la ministre. Autre totem exubérant : les repas végétariens hebdomadaires dans les cantines, dont la généralisation a été supprimée par le Sénat. Le syndicat Culture Viande nous explique que 70 % du poulet servi dans les cantines sont importés de l'étranger, mais tant pis si nos écoliers sont nourris avec de la viande brésilienne : l'important, c'est qu'ils mangent un menu végétarien par semaine ! Sans nouveauté, on constate surtout à quel point la question cruciale de l'environnement est instrumentalisée par des idéologues, qui parlent de planter des arbres, mais s'acharnent surtout à couper nos racines. Cela suffit ! Pour oeuvrer en faveur de l'environnement, nous devons protéger nos producteurs locaux, favoriser les circuits courts, revoir notre place dans la mondialisation. L'écologie ne s'impose pas selon les codes d'un exercice bureaucratique. Cette responsabilité s'exerce localement, dans le quotidien de chacun. Je pense d'ailleurs qu'il existe encore un bon sens local, puisque je ne vois toujours aucune éolienne de 150 mètres de haut dans le jardin du Luxembourg ni de panneaux solaires sur le toit du Sénat Comme alternative à la mondialisation écologiquement désastreuse, nous proposons une écologie de la vie, enracinée et locale, incitative, respectueuse de l'homme et de l'intégrité, notamment visuelle, de la biodiversité. En vue d'y contribuer, je voterai les modifications positives apportées par les sénateurs, portant la parole des élus locaux sur ce projet de loi.

j'avais exprimé notre regret face au manque d'ambition de ce texte non seulement au regard de la volonté affichée et des engagements pris par le Président de la République devant la Convention citoyenne pour le climat, mais aussi du décalage avec le projet de loi de révision constitutionnelle, qui vise à placer au plus haut la question environnementale. Avec d'autres groupes, nous avons rédigé et voté un amendement tendant à imposer à la France de respecter la trajectoire définie par les accords de Paris et la future répartition des efforts négociée au niveau européen en termes d'émissions de CO2. Il s'agissait tout simplement de rappeler au Gouvernement ses obligations, alors que de nombreux observateurs et acteurs- Haut Conseil pour le climat, organisations non gouvernementales (ONG) et parlementaires -s'inquiètent. Plusieurs milliers d'amendements et des dizaines d'heures de débat plus tard,

nous l'avons constaté au cours des débats ou encore à l'instant même, à travers les interventions des orateurs qui m'ont précédé. Cela signifie sans doute que la voie empruntée est la bonne, avec du bon sens et du pragmatisme, sans idéologie ni dogme. J'en veux pour preuve les avancées à tous les titres affichage environnemental, encadrement de la publicité, certification de la neutralité carbone, impact des livraisons, économie sociale et solidaire, commande publique, cycle de vie, pollution des eaux et continuité écologique, forêt,

rénovation performante des bâtiments, pollution des sols, catastrophes naturelles, restauration collective, produits locaux et de qualité, souveraineté alimentaire, déforestation importée ... Cette liste n'est pas exhaustive.

nous ne faisons qu'accompagner la prise de conscience et les réalisations de tous les acteurs engagés- associations, entreprises, agriculteurs, collectivités locales, fédérations syndicats professionnels. Chaque jour qui passe apporte son lot de nouvelles encourageantes : une économie qui se dirige à grands pas vers la décarbonation, le glissement des énergies fossiles vers les énergies renouvelables, des investissements vertueux et responsables De façon irréversible, les enjeux « climat » sont désormais intégrés à tous les niveaux de la société et par chacun de nos concitoyens- je m'en réjouis. Engagé sur ces sujets depuis toujours, je peux attester de cette évolution rapide et positive. Restons lucides cependant : beaucoup reste à faire pour modifier la trajectoire. Mais nous sommes confiants en la capacité de l'homme à accélérer le mouvement amorcé depuis plusieurs années. Nous ne souhaitons pas céder au catastrophisme ou au déclinisme de certains, parce que nous avons intimement besoin d'une « Espérance ». Je crois en l'instinct de survie de notre espèce. Nous saurons ensemble protéger le vivant et faire preuve d'altruisme. J'ai foi en notre humanité.

une fois de plus, le Sénat est arrivé au bout d'un projet de loi « XXL » en y apportant sa touche territoriale. Plus de 4 200 amendements ont été discutés, des dizaines d'articles ont été ajoutés ou réécrits, en commission et en séance publique.

Si l'on en croit les discours indignés des adeptes de la décroissance, le Gouvernement aurait déçu les ambitions de la Convention citoyenne pour le climat. Je pense plutôt que le politique a été suffisamment pragmatique pour ne pas reprendre sans filtre toutes les mesures, de bon sens ou non, élaborées par les « 150 ». En se plongeant dans les centaines de pages du dispositif législatif, un autre diagnostic s'impose : la bien-pensance et la bureaucratie ont trouvé de nombreux terrains d'entente. Il faut le dire clairement : ce texte est une mine d'or pour tous les administrateurs convaincus que la complexification des normes et l'alourdissement des charges sont les gages d'une action publique vertueuse. Bien naïf qui croirait que de simples citoyens, confrontés tous les jours à une administration tatillonne, ont pu élaborer des solutions si complexes et si procédurières aux problèmes climatiques sans l'aide bienveillante des fonctionnaires de l'hôtel de Roquelaure.

Mais, de manière récurrente, nous avons eu l'impression de passer à côté de sujets primordiaux. Comment fixer un objectif ambitieux de diminution des émissions de gaz à effet de serre sans se pencher d'un peu plus près sur l'avenir de notre mix énergétique et en se contentant d'évoquer du bout des lèvres la question du nucléaire ?

alliant des rémunérations dignes de ce nom aux impératifs écologiques. Il faut absolument trouver un consensus dans ce domaine. Arrêtons les surtranspositions et l'autoflagellation Sachons reconnaître que notre agriculture est l'une des plus propres et l'une des meilleures du monde. À écouter les intégristes en tout genre, nous finirons par importer n'importe quoi en matière d'alimentation. De même, nous avons soutenu le développement des bioliquides et des biocarburants, ainsi que le stockage dans le secteur des énergies renouvelables. Ce sont là autant de sujets essentiels pour l'avenir de la France et même de la planète. Malgré la densité de ce texte, je tiens à revenir sur quelques sujets majeurs dont notre attention ne doit pas être détournée. La question de l'énergie nucléaire n'a été qu'effleurée. Or nous pensons que le nucléaire est essentiel à notre bouquet énergétique ... Très bien ! ..., qu'il sécurise notre approvisionnement et que la France doit continuer à innover dans ce domaine.

a fait l'objet de discussions intéressantes. En tant que membre du Conservatoire du littoral, j'insiste une nouvelle fois sur l'extraordinaire importance de celui-ci pour l'ensemble du territoire national. Sa protection est notre devoir, tant sa place pour la préservation de la biodiversité et l'équilibre des espèces est primordiale. Le volet « transports » a été un sujet de réflexions particulièrement intenses. Arrêtons de pénaliser nos propres PME dans le secteur du transport routier de marchandises : il est important de leur donner le temps nécessaire à la transition tout en les accompagnant réellement. Notre transition doit nous permettre de rester compétitifs : elle ne doit pas détruire nos emplois et notre système économique. Très bien ! Enfin, la stratégie nationale de lutte contre l'artificialisation des sols part, le manque de réalisme que traduit parfois ce texte et, d'autre part, l'écart entre l'objectif affiché et les moyens déployés pour l'atteindre. Pas un seul Français ne se réjouit que notre pays se bétonne à vue d'oeil mais aucun ne comprendrait que son logement ou son emploi soit soumis à l'application très stricte de règles émises depuis Paris. Sur ce sujet encore, le Sénat a été force de proposition pour assouplir la mise en oeuvre territoriale de la stratégie nationale. nationale. Nous imaginons à peine les contraintes que ce texte risque de faire peser sur le développement de nos territoires, et tout particulièrement de la ruralité, dans les années à venir. Surtout, nous risquons de leur imposer une double peine : non seulement nous les contraindrons dans leur développement, mais nous pénaliserons davantage les territoires vertueux, qui ont peu artificialisé au cours des dernières années. Les élus de notre groupe ont formulé des propositions afin d'apporter des solutions à ces problèmes.

Le dérèglement climatique est une réalité de tous les jours dans nos territoires, dans le mien, dans le vôtre. Chaque saison se modifie, les sécheresses s'accentuent, les pluies sont désormais diluviennes et nous devons nous adapter rapidement. Mais on ne mènera pas cette adaptation en reculant : c'est pourquoi nous devons trouver des solutions ambitieuses, audacieuses et novatrices.

est certainement perfectible, et nous devrons en tirer des leçons, mais elle a eu le mérite d'essayer de répondre au désarroi d'un certain nombre de nos concitoyens qui souhaitent

chacun a fait sa part du travail et la démocratie représentative a joué son rôle, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Vous

est reprise. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant lutte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 L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement

Il s'agissait, en 2017, de sortir de l'état d'urgence, qui n'avait pas vocation à constituer un état permanent. Il s'agissait aussi de maintenir un niveau extrêmement exigeant de sécurité pour les Français, dans un contexte marqué par une menace terroriste À cette fin, la loi SILT, entrée en vigueur le 1 novembre 2017, a permis le déploiement d'outils nouveaux, mais adaptés, garantissant un équilibre entre efficacité de l'action antiterroriste et préservation des libertés.

Il s'agit pour nous d'amplifier les moyens de la lutte antiterroriste tout en renforçant les garanties entourant la mise en oeuvre des dispositifs opérationnels, dans le strict respect des principes constitutionnels. La mobilisation du Gouvernement pour lutter contre le terrorisme est constante. Depuis 2017, et à la demande du Président de la République, le Gouvernement a oeuvré avec une très grande détermination au renforcement des dispositifs de lutte contre la menace terroriste. Nous l'avons fait en continuant, avec le soutien du Parlement, à augmenter les moyens mis à la disposition des services spécialisés dans la lutte antiterroriste, notamment les services de renseignement. Au total, 1 000 postes y ont été créés depuis 2017. En parallèle, les budgets d'investissement et de fonctionnement des services ont fait l'objet d'un effort financier sans précédent. la lutte contre le terrorisme exige de nous une mobilisation totale. Sous l'autorité du Président de la République et du Premier ministre, avec l'engagement de l'ensemble des forces de sécurité et des services de renseignement, avec l'appui de la justice, nous menons ce combat sans relâche. Nous ne renoncerons jamais à traquer ces ennemis de la République, qui attaquent par la terreur notre mode de vie et nos valeurs : la laïcité, la liberté d'expression, la liberté de conscience- Respect de l'équilibre initial, recherche du plus large consensus, efficacité opérationnelle, détermination dans la lutte contre le terrorisme : tel est le sens du texte qui vous est soumis aujourd'hui. Ce projet de loi n'est pas un point de bascule, bien au contraire : il s'inscrit dans une dynamique dont nous vous avons régulièrement rendu compte. À cet égard, je tiens à saluer les membres de nos services de renseignement, nos policiers et nos gendarmes, qui, chaque jour, accomplissent un travail exceptionnel pour identifier les menaces, suivre les individus dangereux et mettre en échec leurs projets meurtriers.

Dans le même temps, 36 attentats ont été déjoués par nos services, dont 3 encore en 2021. Grâce à la loi SILT, ces services ont continué à disposer, après la fin de l'état d'urgence, d'un cadre législatif efficace et adapté à leur action. L'autorité administrative- préfet ou ministre de l'intérieur selon les cas -s'est vue reconnaître des compétences nouvelles,

de procéder à la fermeture des lieux de culte où se tiennent ou circulent des propos ou théories incitant à la commission ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme ; d'édicter, à l'encontre d'individus présentant un niveau de menace caractérisée pour la sécurité et l'ordre publics,

75 d'entre elles sont actives à ce jour. Enfin, 482 visites domiciliaires ont été réalisées, dont 305 depuis l'attentat contre Samuel Paty, et 256 été effectuées. Ces mesures ont toujours été utilisées de manière ciblée, sous le contrôle du juge. Le Parlement a bien été informé sans délai de la mise en oeuvre de chacune de ces mesures, conformément aux exigences fixées par le législateur en 2017. en 2017. Il a également été rendu destinataire, chaque année, d'un rapport d'évaluation sur la mise en oeuvre de la loi. De la même manière, le Gouvernement a fait un usage raisonné de la technique dite « de l'algorithme ». Ainsi, depuis 2015, trois traitements automatisés ont été autorisés par le Premier ministre, après avis favorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement,

permis de détecter des contacts entre des individus porteurs d'une menace terroriste- il s'agit là d'un point fondamental ; d'obtenir des informations sur la localisation d'individus en lien avec cette menace ; de mettre au jour les comportements de personnes connues des services de renseignement et exigeant des investigations plus approfondies

à donner à la loi SILT. Je le rappelle à mon tour : faute d'intervention du législateur, plusieurs dispositions du code de la sécurité intérieure arrivent à échéance en 2021, après avoir été prorogées de sept mois par la loi du 24 décembre 2020. concernées les dispositions introduites par la loi SILT pour prendre le relais du régime de l'état d'urgence, à commencer par les articles 1 à 4 de ce texte, qui ont instauré des mesures de police administrative inspirées de l'état d'urgence : périmètres de protection, fermeture des lieux de culte, mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, visites domiciliaires et saisies. s'agit de mesures fortement attentatoires aux libertés, le législateur a prévu un contrôle parlementaire renforcé, ainsi qu'une date de caducité de ces dispositions. Initialement fixé au 31 décembre 2020, ce terme a été reporté au 31 juillet 2021. le projet de loi que nous examinons aujourd'hui procède à divers ajustements. Il limite la durée de mise en place des périmètres de protection, élargit la mesure de fermeture administrative des lieux de culte en permettant la fermeture des locaux annexes autorise la saisie des supports informatiques lorsque, à l'occasion d'une visite domiciliaire, la personne fait obstacle à l'accès aux données concernées ou à leur copie. Pour ce qui concerne les Micas, ce projet de loi donne notamment au ministre de l'intérieur le

Face à cet enjeu, le Parlement a adopté, le 27 juillet 2020, une loi instaurant des mesures de sûreté, qui visait avant tout à introduire une nouvelle mesure judiciaire de suivi et de surveillance post-sentencielle. Le Conseil constitutionnel, saisi, a toutefois jugé que la mesure envisagée n'était ni adaptée ni proportionnée et l'a donc déclarée inconstitutionnelle. Nous sommes d'accord sur le constat

qui concerne enfin l'article 18, qui encadre la possibilité pour les services de l'État d'utiliser un dispositif de brouillage des ondes émises par des drones malveillants, il nous a semblé que la base légale proposée était tout à fait pertinente.

Mme Iliana Iotova, vice-présidente de la République de Bulgarie, et de Son Excellence M. Nikolay Milkov, ambassadeur de Bulgarie. En visite en France, Mme Iliana Iotova a été reçue cette après-midi par le groupe d'amitié France-Bulgarie. Elle est accompagnée par notre collègue Loïc Hervé, qui est le président

été encore renforcés par l'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne et à la communauté francophone, dans laquelle elle prend une part active. Nos deux groupes d'amitié travaillent ensemble à une relation toujours plus proche entre le Sénat et le Parlement bulgare. Qu'ils soient assurés de notre plein soutien. Mes chers collègues, en votre nom à tous, permettez-moi de souhaiter à Mme Iliana Iotova la plus cordiale bienvenue au Sénat de la République française ! Nous reprenons

essentiels à la défense de notre souveraineté, et la protection des droits et libertés constitutionnels, au premier rang desquels se situe la protection de la vie privée. Six ans plus tard, il convient de consolider cet équilibre, afin de faire face à une double évolution celle de la menace qui pèse sur la sécurité intérieure et la défense de notre pays ; d'autre part, celle qui est liée à l'essor des nouvelles technologies. Les derniers attentats, ceux de Conflans-Sainte-Honorine et de Rambouillet ont montré que le risque terroriste évoluait vers un « djihadisme d'atmosphère », comme le qualifie Gilles Kepel, nécessitant de nouvelles méthodes pour détecter les « signaux faibles » du passage à l'acte. S'y ajoute une menace exogène persistante et la montée en puissance de certaines mouvances contestataires, l'exacerbation d'actions subversives violentes. Par ailleurs, les nouvelles techniques de communication, comme la 5G ou les communications satellitaires, imposent de doter les services de la communauté du renseignement français des moyens adaptés à l'évolution des pratiques des terroristes et des criminels.

Limité à la finalité de la lutte contre le terrorisme, le traitement automatisé des données de connexion a montré tout son potentiel. C'est pourquoi nous vous proposerons de pérenniser cette technique dans son principe,

L'autre menace juridique qui pèse sur les techniques de renseignement provient directement de l'application des normes européennes ! L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 octobre 2020, ainsi que celui du Conseil d'État,, qui en tire les conséquences, fragilise le système de conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic et de localisation. Les articles 15 et 16 du projet de loi, profitant du « chemin de crête » tracé par le Conseil d'État, précisent et encadrent la conservation de ces données.

en cas d'infractions pénales ordinaires, je vous propose d'adopter ces articles qui maintiennent les capacités opérationnelles des services de renseignement. Néanmoins, afin d'en atténuer l'impact, je vous soumettrai un amendement visant à préciser que les données de trafic et de localisation peuvent être utilisées pour la recherche des auteurs d'actes de criminalité et de délinquance grave. Le corollaire de l'extension des moyens des services de renseignement est le renforcement du contrôle. Le secret qui entoure naturellement le travail quotidien des agents des services de renseignement, auquel je veux rendre hommage pour leur dévouement et pour la protection qu'ils nous garantissent, est souvent source de fantasmes.

à la difficile question de l'accès aux archives intéressant la défense nationale, elle a fait l'objet d'échanges nombreux entre les commissions des lois, de la défense et des affaires culturelles du Sénat.

serait de nature à nuire aux intérêts fondamentaux de la Nation. À condition- nous y insisterons -que les services détenteurs de ces documents sensibles fassent leur inventaire dans des délais raccourcis, l'équilibre entre la protection du secret-défense et le libre accès aux archives est, selon nous, assuré par ce texte.

Ces articles concernent les services de renseignement, les techniques d'investigation qu'ils peuvent utiliser, la lutte contre les drones présentant une menace, ainsi que les archives intéressant la défense nationale. Le contexte sécuritaire national reste marqué par le terrorisme, et le continuum sécurité-défense constitue toujours un enjeu crucial pour la sécurité de nos concitoyens, quoique la menace soit plus endogène que par le passé. Nos armées affrontent sans relâche une menace terroriste globale. La fin annoncée de Barkhane, sur laquelle nous aurions aimé avoir des indications lors du débat qui a eu lieu ici même, ne signifie

le terrorisme constitue la première des menaces, nos services ne cessent de faire face également aux agissements de puissances étrangères de plus en plus décomplexées, qui utilisent tous les moyens fournis par les nouvelles technologies et par le cyber. Dans ce contexte, il était important que les services de renseignement, ceux du ministère des armées comme ceux des autres ministères, continuent de disposer des moyens les plus efficaces et les plus performants pour mener leur action. La création d'un régime des interceptions satellitaires, la possibilité de solliciter les opérateurs de télécommunications en matière d', afin de s'adapter à la 5G, ou encore l'extension des algorithmes aux URL, permettront ainsi aux services de rester dans la course technologique. Par ailleurs, nous nous félicitons de la possibilité nouvelle de brouiller les drones menaçants. En effet, cette menace est loin d'être théorique. La gendarmerie nationale est d'ailleurs en pointe sur ce sujet. Il fallait en outre, pour encadrer cette évolution, des règles juridiques répondant à deux nécessités : premièrement, la continuité avec le cadre fixé par la loi du 24 juillet 2015, car les services ont formé leurs agents à ce cadre et ont désormais besoin de stabilité deuxièmement, des garanties suffisantes pour que les libertés, en particulier la vie privée, ne subissent pas d'atteinte excessive. Le projet de loi, nous semble-t-il, répond bien à ces deux exigences, et les modifications introduites par la commission des lois consolident encore cet équilibre. Concernant les interceptions satellitaires, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a souhaité, en concertation avec la commission des lois, restreindre l'expérimentation aux services du premier cercle. Il s'agit en effet d'une technologie à large spectre et pour le moment très expérimentale ; d'où la nécessité d'encadrer et de centraliser son usage autant que possible. Il sera toujours temps ensuite de l'ouvrir à d'autres services- je pense en particulier à la gendarmerie nationale, qui pourrait à l'avenir Grâce aux amendements adoptés à l'Assemblée nationale, le projet de loi renforce par ailleurs les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement, la DPR. Ainsi se trouve conservée la proportionnalité entre les pouvoirs des services et l'étendue du contrôle parlementaire, qui constitue un élément clé de notre système.

spéciaux, la CVFS. Quant au nouveau régime de communication des archives, enfin, nous avons conscience qu'il suscite des débats, mais l'équilibre atteint nous semble solide. Je rappelle notamment que le réexamen des délais de communicabilité est très fréquent dans les services d'archives.

La modification des informations relatives à la communicabilité de documents d'archives s'effectue désormais en temps réel et toujours au profit de l'usager. Sous réserve de ces remarques et des amendements qui ont été adoptés par la commission des lois lors de l'élaboration de son texte, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a approuvé le présent projet de loi. La parole est à M. le rapporteur

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous devons à la Révolution française le principe selon lequel les archives, leur gestion et leur communication sont des éléments constitutifs de l'État de droit, de la citoyenneté démocratique et de la construction de la mémoire de la Nation. Dans un rapport rendu au Premier ministre en 1996, Guy Braibant décrivait ainsi ces relations : « Il n'y a pas d'Histoire sans archives [ ...] ; il n'y a pas d'Administration sans archives [ ...] ; il n'y a pas de République sans archives. de ces sages principes a toujours été empêchée par les réticences, les obstructions et les dissimulations d'administrations qui se considéraient comme les seules propriétaires des actes publics qu'elles produisaient et qui s'arrogeaient la licence de décider de leur publicité. Les lois de 1978 sur l'accès aux documents administratifs et de 1979 sur les archives ont eu pour objet d'organiser les droits des citoyens à connaître de leur administration au présent et dans le temps.

Cette loi de 2008 réaffirme le principe fondamental de la libre communication des archives publiques, auquel ne peuvent être opposées que des dérogations consenties et garanties par le législateur. Dans la pratique, elle confère au ministère de la culture une mission interministérielle de coordination, de contrôle et de promotion des politiques publiques des archives. Cet édifice législatif a été ébranlé en 2011 et en 2020 par deux instructions générales interministérielles qui ont imposé, sous la forme administrative subalterne de l'arrêté, la prééminence du code pénal sur le code du patrimoine et qui ont organisé l'incommunicabilité de documents produits voilà plus de cinquante parce qu'ils étaient classés au titre du secret de la défense nationale. Ainsi, des documents qui étaient librement disponibles ont dû faire l'objet de procédures de déclassification pour être de nouveau accessibles.

Néanmoins, il considère que, exceptionnellement, les administrations peuvent ne pas autoriser leur divulgation quand celle-ci représente « une menace grave pour la sécurité nationale Comme le rapporteur du Conseil d'État, je regrette que des moyens humains très considérables aient été consacrés à la déclassification d'environ un million de pièces, que des travaux d'historiens aient été entravés et que des domaines entiers de la recherche historique aient été délaissés à la suite d'une analyse juridique aussi peu assurée.

l'article 19, qui institue un nouveau régime dérogatoire pour certains des documents déjà soumis au délai d'incommunicabilité de cinquante ans. Peut-être eût-il été de bonne politique d'attendre la décision du Conseil d'État et de ne pas légiférer dans l'extrême urgence alors que le rapporteur public considère que l'administration peut toujours appliquer les dispositions du code du patrimoine « à la lumière de l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation Par ailleurs, notre commission regrette que le Conseil supérieur des archives et la Commission d'accès aux documents administratifs n'aient pas été consultés sur cette révision importante de la loi de 2008. À l'unanimité de ses membres, la commission de la culture du Sénat a exprimé ses fortes réticences à voter en l'état un article qui révise le principe de la loi de 2008 en faisant porter sur les lecteurs et les services des archives la charge de la détermination de la communicabilité des documents. La commission de la culture a formulé plusieurs propositions, dans le respect du principe constitutionnel de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, pour que les administrations réalisent le récolement de leurs fonds en fonction des nouvelles normes de communication et en informent les usagers des archives.

le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires tient tout d'abord à affirmer, face au présent texte, son sentiment premier, à savoir une grande inquiétude. Nous remarquons en effet que, depuis quelques années maintenant, la France est le théâtre d'une succession de lois sécuritaires, qui se veulent antiterroristes, mais qui sont surtout liberticides.

petit bout par petit bout, les libertés individuelles des Français. Oui, lutter efficacement contre la menace terroriste est un objectif que nous visons tous. Mais cela ne peut se faire au prix de l'affaiblissement des droits et libertés garantis par notre Constitution. Cette longue suite de textes liberticides aboutit aujourd'hui à ce projet de loi. Venons-en donc aux faits. La présente motion vise à déclarer irrecevable le projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement en raison des risques d'irrecevabilité constitutionnelle que présentent certaines de ses dispositions portant atteinte à la liberté

autant de libertés que nous nous devons, nous, législateurs, de ne pas mettre en péril par la loi. En premier lieu, ce projet de loi reprend, dans son article 5, des dispositions précédemment censurées par le Conseil constitutionnel. En effet, la loi n° 2020-1023 du 10 août 2020, dite « Mesures de sûreté », a fait l'objet d'une large censure de la part du juge constitutionnel dans sa décision n° 2020-805 DC

à la liberté d'aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale d'une manière que le Parlement introduise de nouveau dans un projet de loi une disposition précédemment jugée attentatoire aux libertés individuelles et écartée par le Conseil constitutionnel.

l'assignation à résidence, les périmètres de protection. La récurrence des états d'urgence, la prorogation de ces mesures, puis leur pérennisation, ont pour effet de limiter nos libertés publiques individuelles des impératifs de sécurité de nos concitoyens. Mais que protègent-elles réellement, ces mesures qui affaiblissent tant les libertés des Français ? Le recours intensif à des procédures administratives, jugées plus rapides que les procédures judiciaires, doit nous alerter : de telles procédures contournent le contrôle du juge judiciaire, garant des libertés individuelles conformément à l'article 66 de la Constitution. Cette déjudiciarisation en marche doit, là encore, sérieusement nous alerter. En troisième lieu, la surveillance généralisée des URL prévue aux articles 13 et 14 porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, pourtant reconnu comme principe à valeur constitutionnelle depuis la décision n° 99-416 DC du Conseil constitutionnel en date du 23 juillet 1999. la CNIL, estime en ce sens que le recueil des URL est susceptible de faire apparaître des informations relatives au contenu des éléments consultés ou aux correspondances échangées. Sur l'ensemble des dispositifs qui concernent le déploiement des mesures de renseignement,

Le Premier ministre peut ainsi toujours déroger à l'avis de cette commission, ce qui nous semble problématique. équilibre entre la sécurité publique, la protection des intérêts fondamentaux de la Nation et le respect de la vie privée nécessite des garanties, ainsi que le contrôle par une autorité indépendante du pouvoir politique. Enfin, les restrictions à l'accès aux archives prévues à l'article 19 du présent texte contreviennent au droit d'accès aux documents administratifs, pourtant consacré

Ce projet de loi avait initialement pour objet de renforcer l'arsenal pénal pour répondre à l'enjeu sécuritaire du terrorisme. Mais il perd de vue cet objet et tombe dans le piège où ont les précédentes lois attentatoires aux libertés individuelles. Comme nous le déplorons régulièrement devant ce type de textes, force est de constater qu'aucune réflexion de fond n'est encore menée quant au problème réel que représente la radicalisation, particulièrement en détention. Face à la menace terroriste, la réponse législative se démultiplie, au rythme de plus d'une loi par an depuis dix ans. L'efficacité des dispositifs votés est parfois hypothétique, alors qu'ils rognent sans ménagement les libertés fondamentales. Cette accumulation de lois sécuritaires

de vue de son efficience en matière de réduction du risque terroriste. L'objectif politique est manifestement de « cranter » les thématiques régaliennes avant la présidentielle, la sécurité étant devenue un thème omniprésent dans le débat public. Inscrire dans notre droit commun des procédures d'exception affaiblit peu à peu notre État de droit ; nous ne saurions en être complices. Ainsi, en application de l'article 44, alinéa 2, du règlement, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires invite le Sénat à déclarer irrecevable le projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, adopté par la commission des lois le 16 juin 2021. Personne ne

Monsieur le président, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, au préalable, je souhaite être très claire sur un point le Gouvernement et la majorité sénatoriale de droite n'ont pas le monopole du souci de la sécurité, comme nous n'avons pas, à gauche, celui de la protection des libertés. Tâchons de ne pas considérer ceux qui critiquent le texte comme des ennemis de la sécurité et ceux qui ne souhaitent pas l'améliorer comme des ennemis de la liberté ! Qui ne souhaite pas prévenir les actes de terrorisme dans notre pays ? Personne. Il est nécessaire de rappeler ici que les crimes odieux qui nous ont endeuillés ces dernières années en France sont des actes commis pour la quasi-totalité au nom d'un islamisme politique qui alimente la peur et attise la haine de l'autre pour propager les idéologies les plus mortifères.

Dans ce cadre, et en parallèle à l'action nécessaire à mener, il est de la responsabilité du politique, et plus encore des acteurs issus de la gauche progressiste, de se montrer rassurant, en réaffirmant certaines valeurs et en éclairant les débats. Il m'est aujourd'hui difficile de constater que, s'agissant de certains débats politiques, ma formation est contrainte d'expliquer en quoi les idées progressistes qui l'animent sont à l'exact opposé de cet obscurantisme au service duquel évoluent les terroristes qui portent atteinte à notre Nation. Mes chers collègues, madame la ministre, nous partageons la même intransigeance issue du même constat : nos concitoyennes et nos concitoyens ont le droit de vivre en paix sur notre territoire.

les attentats diffus que nous connaissons ces dernières années ne sont-ils pas, pour certains, des passages à l'acte d'individus dont la folie se cristallise sur la haine de l'autre que véhicule le terrorisme islamiste ? Un début de réponse à ce phénomène est amorcé avec l'article 6 de ce projet de loi mettant en oeuvre une perméabilité dans la communication des informations sur des individus faisant l'objet de mesures de soins psychiatriques sans consentement. Cette extension du nombre de personnes ayant accès à une information médicale contrevient au principe du droit au respect à la vie privée et au secret des informations médicales. comme le dénoncent des syndicats, parmi lesquels le Syndicat de la magistrature, « ces dispositions ne font finalement qu'entériner des pratiques d'un autre âge reposant sur l'idée qu'un fou est par nature dangereux Si, selon vous, cette nouvelle menace diffuse doit aboutir à un système de surveillance et de répression plus fin, plus complet et plus dur, cela nous semble, pour notre part, être un leurre, d'abord, parce qu'il sert le modèle de ceux qui réfutent notre État de droit, ensuite, parce que ce système est inefficace. Concernant les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, les Micas, que vous souhaitez pérenniser, au moment de leur mise en oeuvre et des premiers débats parlementaires, l'ancien juge antiterroriste, Marc Trévidic, s'exprimait en ces termes : « Face

en quoi ils sont moins dangereux ensuite ? Tout homme sensé comprend que l'on attise le feu avec de telles méthodes. On tape n'importe qui, n'importe comment. » Comme l'ont illustré les travaux de la commission des lois du Sénat, qui s'est attachée une fois de plus à un rôle de correctrice de la loi, le texte présenté par le Gouvernement avait la particularité de cumuler un nombre remarquable de risques d'inconstitutionnalités. Sur les mesures administratives, pourquoi le Gouvernement persiste-t-il, notamment, à porter la durée maximale des Micas de douze à vingt-quatre mois, alors même que le Conseil d'État n'a pas retenu cette disposition, estimant qu'elle soulève une difficulté d'ordre constitutionnel, sans que son efficacité soit suffisamment établie Une inconstitutionnalité plus lourde encore pèse sur les mesures de sûreté : le Gouvernement a repris à son compte, sous un habillage de réinsertion, le dispositif porté par Yaël Braun-Pivet, lequel avait été censuré presque intégralement par le Conseil constitutionnel en août 2020.

Aucune de ces réécritures ne nous convainc, puisque l'économie générale des dispositifs est conservée et porte atteinte à notre État de droit, en cherchant à aiguiser davantage notre arsenal répressif par de douteux motifs visant la dangerosité supposée de certains individus ayant déjà purgé leur peine,

réduisant au maximum les remises de peine et conduisant finalement à un problème de sorties sèches. C'est ce problème que vous cherchez à résoudre depuis maintenant plus d'un an, et vous semblez être dans l'impasse. En effet, une fois la peine purgée, que faire de ces personnes ? Instaurer une sorte de peine après la peine avec les nombreuses mesures de sûreté que vous souhaitez mettre en oeuvre, c'est faire l'aveu de l'échec de notre système pénitentiaire et du traitement de ces condamnés. De la détention au suivi post-carcéral, en passant par la répression, rien, dans le système que vous venez consolider, ne peut éviter actes de terrorisme ou récidives. En outre, le système de pseudo-prévention que vous imaginez n'est ni efficient ni souhaitable pour notre démocratie.

tout en maintenant à distance l'autorité judiciaire. Avec l'ensemble de ces techniques, le Gouvernement se dote d'un arsenal de surveillance de masse.

que la technique ne serait pas politique. En effet, la technique est bien politique, et il convient de remettre le débat sur le terrain des valeurs. La lutte contre le terrorisme ne sera efficace et effective que lorsque nous commencerons par traiter non ses symptômes, mais ses causes. De nombreuses questions restent, selon nous, en suspens pour traiter sérieusement le sujet. Quel bilan tirons-nous de toutes les lois antiterroristes votées ces dernières années ? Leur échec flagrant ne doit-il pas nous inviter à revisiter la méthode engagée ? La prévention ne devrait-elle pas prendre le pas sur la répression, la déflation carcérale sur l'inflation carcérale la police de proximité, de prévention et de dissuasion sur la police uniquement répressive ? Nous répétons inlassablement notre attachement à ce modèle de police républicaine, car nous sommes persuadés que le renseignement français sortirait grandi d'une coopération renforcée avec des policiers, au plus proche de nos concitoyens. Enfin, au niveau diplomatique, ne faudrait-il pas cesser tout échange avec des pays dont l'attitude envers les factions terroristes est parfois trouble ? À jeter en pâture nos libertés publiques, notre pays ne sortira pas grandi, et notre sécurité collective ne se trouvera aucunement renforcée. Ce que veulent nos ennemis obscurantistes, c'est le recul de nos démocraties, la mise à mal de nos droits et de nos libertés publiques, pour revenir à cet état primitif de la loi du plus fort. La France doit se ressaisir et rester fidèle aux idéaux qu'elle porte depuis le siècle des Lumières, en renonçant au chemin de la surenchère sécuritaire.

le 31 juillet 2021. Ces mesures de police administrative ont fait la preuve de leur efficacité, et nous sommes dans l'obligation de les inscrire dans la loi. La deuxième raison repose sur le fait que la commission des lois

et que nous entendons soutenir avec ferveur et détermination en séance. C'est, en particulier, le cas du dispositif de suivi des personnes condamnées pour des actes terrorisme ayant purgé leur peine, initialement proposé par notre président François-Noël Buffet. Chacun ici peut mesurer l'importance et la portée La troisième et dernière raison tient à l'exigence de donner aux différents acteurs de la communauté du renseignement les moyens de lutter efficacement contre les menaces renouvelées ou émergentes auxquelles notre pays doit faire face demain et dans les années à venir. Pour l'ensemble de ces raisons, notre groupe votera contre la motion tendant à opposer la question préalable présentée par nos collègues communistes.

mais de fond, préparé depuis plusieurs mois et élaboré à partir d'une double nécessité. D'une part, il s'agit de l'échéance prochaine de cinq mesures, auxquelles il avait été conféré un caractère expérimental au sein de la loi Renseignement de 2015 et de la loi SILT de 2017 et dont le terme a été repoussé par l'adoption d'une loi à la fin de l'année dernière. D'autre part, ces mesures sont utiles pour faire face à une menace terroriste persistant à un niveau élevé sur le territoire national et présentant un caractère endogène et évolutif. Cet état de fait impose que les services de renseignement et les forces de sécurité disposent de moyens opérationnels et d'un cadre juridique adapté à la réalisation de leurs missions, notamment au regard des évolutions et des usages technologiques.

des atteintes à l'ordre public et respect des droits et des libertés. Le projet de loi opère à ce titre plusieurs choix opportuns, dont certains suscitent une convergence dans cet hémicycle. Il propose tout d'abord de pérenniser les cinq mesures précitées au regard de leur utilité démontrée et de leur mise en oeuvre équilibrée, relevée notamment dans les rapports d'information parlementaires, dont celui de la mission pluraliste de la Haute Assemblée.

le cas de la technique expérimentale de captation des communications satellitaires, de l'extension aux URL de la technique des algorithmes pour détecter les signaux faibles, ou encore de la faculté de recourir à des dispositifs de brouillage radioélectrique à l'encontre de drones présentant une menace.

Cette décision, par les limites qu'elle pose aux États membres, suscite la crainte d'un affaiblissement de nos capacités de lutte contre la délinquance ne relevant pas de la criminalité grave. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de l'examen d'un amendement des rapporteurs qui tend utilement à préciser cette notion. notion. Je m'arrêterai enfin un instant sur un point, au regard des positions qui viennent d'être exprimées en présentation des motions : le texte prévoit d'accroître un certain nombre de garanties en matière de sécurité intérieure et de renseignement, avec le renforcement de l'encadrement des modalités de transmission des informations entre services et aux services de renseignement et celui des garanties procédurales entourant la mise en oeuvre des algorithmes ou encore celui du contrôle de la CNCTR, notamment par la généralisation du caractère suspensif instance. Enfin, il affirme le contrôle parlementaire au travers, notamment, des prérogatives dont jouit la délégation parlementaire au renseignement. L'ensemble de ces garanties affermies, ainsi que les différents dispositifs précités, a été confirmé lors de l'examen en commission, et je salue le travail de nos rapporteurs,

et de la création d'une mesure judiciaire de réinsertion, d'autre part, les rapporteurs préfèrent donc une unique mesure judiciaire intégrant à la fois les finalités de réinsertion et de surveillance. Ces deux propositions concurrentes nous imposent de choisir la moins risquée du point de vue constitutionnel et nous enjoignent donc au parti pris. Au regard de la censure du Conseil constitutionnel intervenue l'été dernier à propos d'une mesure judiciaire comportant un nombre d'obligations proche de la mesure retenue par la commission, il apparaît que le risque constitutionnel existe et pèse également sur cette version. Enfin, nos débats s'achèveront par l'examen du régime de communicabilité des archives classifiées à l'article 19, disposition qui a fait l'objet d'un certain nombre de modifications à l'Assemblée nationale pour en limiter les effets de bord. Au-delà du cadre législatif, il semble important de mener une réflexion qui relève de l'organisation de l'État sur la qualité des personnes qui seront désignées pour apprécier le prolongement, au-delà de cinquante ans, de l'incommunicabilité des documents relevant des exceptions visées par le projet de loi.

Les problématiques liées au terrorisme et, par conséquent, au renseignement, s'inscrivent désormais comme des préoccupations quotidiennes pour nos concitoyens, donc pour de nombreux services administratifs et judiciaires. Naturellement, le législateur s'implique pleinement, lui aussi, dans la lutte contre ce fléau barbare. Dès 2017, la loi SILT était venue introduire de manière temporaire dans notre droit diverses mesures inspirées des dispositions de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. Depuis lors, il nous revient, malheureusement, la tâche de pérenniser ces dispositifs, donc de nous confronter à une difficulté fondamentale : maintenir le respect et l'équilibre entre État de droit et libertés individuelles. Bien entendu, le Conseil constitutionnel est là pour y veiller ; il l'a encore montré récemment dans sa décision du 7 août 2020 par laquelle il a censuré le dispositif adopté par notre Parlement cet été, lequel introduisait une nouvelle mesure judiciaire de suivi, à leur sortie de détention, des individus condamnés pour des faits de terrorisme. Aussi, certaines du projet de loi examiné ce jour répondent à cette censure des juges. Je veux, à ce titre, saluer le travail du Sénat, qui s'est montré particulièrement réactif en adoptant, dès le 25 mai 2021, la proposition de loi renforçant le suivi des condamnés terroristes sortant de détention. Pour faire fructifier efficacement ce travail parlementaire, il est évident que cette proposition doit s'intégrer au nouveau texte

En ce qui concerne le volet « terrorisme », le législateur s'était montré précautionneux lors de l'examen de la loi SILT, en adoptant des mesures temporaires, d'application limitée au 31 décembre 2020. Ce délai a dû être prorogé au 31 juillet 2021, mais il n'était pas possible de reporter cette pérennisation inlassablement, sauf à renoncer à ce que notre droit bénéficie d'une forme de stabilité. Ce projet de loi permet ainsi d'aller au-delà de cette date, en ne retenant plus de limitation dans le temps, avec l'espoir qu'une telle disposition ne soit pas attentatoire aux garanties constitutionnelles exigées. Cependant, les ajustements apportés par notre commission des lois devraient contribuer à atteindre l'équilibre espéré. Je pense en particulier à l'article 1 , qui a été introduit lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale et que la commission a amendé, en intégrant certaines réserves d'interprétation formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 mars 2018. Concernant le volet renseignement, ce projet de loi ajuste ou modifie un certain nombre de mécanismes institués par la loi du 24 juillet 2015. Comme cela a déjà été souligné, il apparaît nécessaire, d'une part, de travailler à un meilleur encadrement de l'exploitation et de la transmission de renseignements entre services et aux services, d'autre part, d'oeuvrer pour adapter les moyens de nos services de renseignement aux nouvelles formes de menaces toujours plus diffuses. Enfin, ce projet de loi aborde un point délicat : la classification des archives. En effet, l'article 19 modifie le régime d'accès aux archives classées secret-défense en allongeant potentiellement au-delà de cinquante ans le délai pendant lequel ces archives peuvent ne pas être accessibles, notamment aux chercheurs, aux historiennes et historiens, et, plus généralement, aux citoyens.

prévoit d'actualiser la loi Renseignement en tenant compte des évolutions technologiques, en particulier la mise en oeuvre prochaine des réseaux téléphoniques par satellite et de la 5G, mais aussi du besoin d'algorithmes traitant les URL. d'améliorer la régulation des échanges entre les services de renseignement et les autres administrations. Le troisième volet tire les conséquences de la décision de la CJUE concernant les

Avant d'entrer dans le détail, je souhaite, au nom du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, saluer la mémoire de ceux qui ont été frappés par le terrorisme au cours des dernières années.

déterminés et fidèles à nos valeurs. Cela suppose des textes clairs, des budgets qui donnent les moyens d'agir, ainsi qu'un cadre respectant les libertés individuelles et les principes de l'État de droit. Telle sera notre boussole au cours de l'examen de ce texte. Votée à l'automne 2017,

Soucieux que notre pays dispose d'un arsenal permettant de faire face, dans le respect du droit, aux risques actuels, nous soutiendrons certaines dispositions de ce texte

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, voici le cinquième texte en cinq mois sur la sécurité intérieure ! Cette inflation législative bien française prouve deux choses

chacun prenant isolément sa part par le petit bout de sa lorgnette, sans vision politique cohérente. En refusant de comprendre la dynamique de l'histoire qui s'applique à notre temps, vous courez après la réalité avec le boulet de l'idéologie du « vivre ensemble » accroché au pied. Mais la réalité s'emballe dans un cycle destructeur, sans que vous puissiez l'arrêter. Souvenons-nous de l'islamiste Mickaël Harpon, qui a égorgé ou poignardé à mort quatre de ses collègues policiers en octobre 2019. Rappelons qu'il était informaticien à la direction des renseignements de la préfecture de police de Paris et qu'il était « habilité secret-défense Si le Gouvernement ne comprend pas le problème global de l'immigration-islamisation, les Français continueront à en payer le prix du sang. Vous nous demandez aujourd'hui d'étendre les prérogatives des services de renseignement, quand eux-mêmes sont gangrénés de l'intérieur par un ennemi infiltré ! Nous pourrons toujours renseigner plus et mieux, mais nous n'arrêterons pas la dynamique d'islamisation tant que celle-ci sera alimentée par une déferlante migratoire, une démographie conquérante et un rejet de notre modèle français. Pour protéger nos compatriotes, notre arsenal de défense et de renseignement doit utiliser des outils modernes. C'est pourquoi je suis favorable à l'interception satellitaire des communications, à l'adaptation à la 5G de l'interception de télécommunications par, à l'extension du champ d'application des algorithmes aux adresses des pages internet et au brouillage des ondes pour la lutte anti-drones. Cependant, moins vous ciblez l'islamisme comme ennemi principal, plus vous retirez de libertés à chaque citoyen. À l'origine exogène à notre France, l'islamisme devient par l'immigration massive et le rejet de toute assimilation une menace endogène. Plus d'immigration, c'est plus d'islamisme, et plus d'islamisme, même sans attentat, c'est moins de libertés. En faisant reculer les libertés de tous, vous ne contraignez nullement ceux qui se mettent en dehors des règles et des lois à s'y soumettre. Dans ce texte, il n'y a toujours rien sur le renforcement des obligations de quitter le territoire français, toujours rien sur le suivi de longue durée des terroristes et des radicalisés et toujours rien sur le fichage des mineurs islamistes. Pourtant, sur ce dernier point, il faut rappeler que les quatre derniers projets d'attentats déjoués par la DGSI depuis la fin octobre 2000 ont tous été fomentés par des individus mineurs de 15 à 17 ans ou ayant tout juste atteint leur dix-huitième anniversaire. Quand on pense que la jeunesse d'aujourd'hui forme le pays de demain, on se demande si capter des URL suffira à faire en sorte que la France reste la France, que la France reste française. Mes chers collègues, puisse cette réflexion générale vous guider pendant l'examen de ce projet de loi, avec une détermination proportionnelle à l'urgence.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, « je ne connais rien de plus servile, de plus méprisable, de plus lâche, de plus borné qu'un terroriste » disait l'auteur des, notre célèbre notre célèbre Chateaubriand. Face aux terroristes, nous devons être d'une détermination sans faille. Le terrorisme menace et frappe notre territoire avec intensité depuis plusieurs années. de rendre hommage à la mémoire de Stéphanie Monfermé, tombée sous les coups d'un islamiste à Rambouillet, ainsi qu'à tous nos compatriotes victimes du terrorisme et à leurs familles. Nous savons que les forces de l'ordre, notamment les services de renseignement, sont pleinement mobilisées, pour lutter tant contre les organisations terroristes que contre ce que l'on appelle « les loups solitaires Cette lutte de tous les instants nécessite des dispositifs et des technologies en perpétuelle évolution. Nombre de ces outils peuvent être attentatoires aux libertés : nous devons donc être particulièrement vigilants quant à leur emploi. Le Parlement a ainsi veillé à encadrer strictement plusieurs mesures récemment introduites dans notre droit, comme les périmètres de protection, la fermeture des lieux de culte ou encore les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, les Micas.

la sécurité de nos concitoyens est une priorité, elle ne doit pas être obtenue en faisant peser une menace sur leurs libertés. La commission du Sénat a eu le courage de proposer une solution d'équilibre pour l'extension du champ de la surveillance aux adresses URL : celles-ci pourront être collectées et traitées tant par les algorithmes de détection que par les recueils de données en temps réel. Un tel traitement permettra aux services non seulement de savoir à quels sites se sont connectés les suspects, mais aussi de connaître les contenus auxquels ceux-ci ont accédé. Ces données donneront un avantage certain aux services de renseignement, mais leur recueil fait peser un risque majeur sur la liberté des Français. C'est pourquoi le Conseil constitutionnel et, après lui, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et la CNIL se sont opposés à leur exploitation. Nous croyons donc qu'il est sage, comme le prévoit le texte voté par la commission, de s'assurer préalablement des conséquences de l'application de ces dispositions, dans le cadre d'une expérimentation temporaire. Le texte prévoit en outre d'autres dispositions destinées à améliorer les capacités de nos services de renseignement, telles que les interceptions de communications satellitaires ou encore l'échange de renseignements entre services, selon une procédure qui en permet la traçabilité. Au-delà de la détection, ce projet de loi introduit également des mesures destinées à prévenir la récidive terroriste et à favoriser la réinsertion. Celles-ci permettront d'assurer sur plusieurs années la prise en charge sanitaire et sociale des personnes condamnées pour terrorisme qui en ont besoin, mais aussi d'améliorer leur suivi. Ces nouvelles possibilités tant techniques que juridiques ne doivent pas nous faire oublier l'essentiel : les moyens financiers sont incontournables. La prévention du terrorisme et de la récidive, la sécurité et la justice sont des sujets essentiels pour nos concitoyens. Les services de l'État, particulièrement lorsqu'ils sont aussi régaliens que les services de sécurité, doivent disposer du budget nécessaire au bon accomplissement de leur mission. Le groupe Les Indépendants - République et Territoires soutiendra donc l'adoption de ce projet de loi, en demandant au Gouvernement de continuer son effort budgétaire dans ces domaines.

Il reprend en effet certaines dispositions de la loi SILT, ainsi que des mesures du régime de l'état d'urgence, telles que la fermeture des lieux de culte, la perquisition administrative ou les saisies informatiques, en prévoyant même un durcissement de certaines d'entre elles.

cette déjudiciarisation en marche suscite une opposition ferme de notre part. Où allons-nous si le principal garde-fou qu'est le juge est de plus en plus souvent dessaisi de sa mission de protection des droits et libertés fondamentales ? Ces mesures administratives, qui constituent l'équivalent des assignations à résidence prises dans le cadre de l'état d'urgence, ne devaient normalement être expérimentées que jusqu'au 31 juillet prochain. Or voilà que le présent projet de loi prévoit leur pérennisation dans notre droit pénal ! Nombre de défenseurs des libertés publiques sonnent l'alarme lorsque de telles mesures temporaires justifiées par une situation de crise sont intégrées dans le droit commun. Cette crainte est légitime : allons-nous instituer une société qui vit dans un état d'urgence permanent ? Ce projet de loi fait également réapparaître les mesures de sûreté judiciaire. Rappelons tout de même que, que, à l'été dernier, le Conseil constitutionnel avait censuré une loi émanant du parti présidentiel qui visait à renforcer les mesures de sûreté prises à l'encontre des détenus condamnés pour des actes terroristes et sortant de prison. Un tel régime d'application rétroactive porte une atteinte excessive aux droits et libertés garantis par la Constitution, alors même que le droit commun prévoit déjà toute une série de mesures permettant d'assurer un suivi post-détention. Enfin, et surtout, ce texte fait courir le grave risque d'une surveillance de masse de la population. Boîtes noires algorithmiques, dispositif, captage des données de communications satellitaires, recueil des URL : tout y est. En 2015, c'était le gouvernement Valls qui avait imaginé un cadre juridique ouvrant la voie aux boîtes noires algorithmiques ... Nous connaissons toutefois les failles de ce système de surveillance. De nombreux spécialistes ont d'ailleurs jugé sévèrement cette initiative. Citons simplement Patrick Calvar, ancien numéro un de la DGSI, qui évoquait dès le début de l'année 2018 la « puissance toute relative des renseignements, même avec des moyens ». Mes chers collègues, nous devons nous poser la question suivante : jusqu'où irons-nous ? Sommes-nous prêts à continuer de réduire, loi sécuritaire après loi sécuritaire, la protection des libertés individuelles des Français ?

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce projet de loi, cela a déjà été dit, intervient à la suite de multiples lois lois sécuritaires dérogatoires au droit commun, votées sans véritable évaluation préalable des dispositifs existants, de leur nécessité ni d'ailleurs de leur efficacité. Il s'agit de pérenniser des dispositifs issus de la loi SILT de 2017, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance. Semblables à des assignations à résidence et à des perquisitions contrôlées par l'administration, ces dispositifs contournent la procédure judiciaire et les droits de la défense et emportent des conséquences particulièrement lourdes pour les personnes visées, jugées sur des motifs d'ailleurs flous de dangerosité. En pérennisant ces mesures, le Gouvernement fait donc le choix d'opérer un tournant radical en matière de police administrative, inspiré par un principe de précaution incompatible avec nos principes démocratiques fondés sur un droit pénal d'interprétation stricte. Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste affirme avec détermination la nécessité de combattre le terrorisme. Notre République doit se doter de moyens à sa hauteur pour assurer un cadre de vie serein sur son territoire, mais cela ne doit en aucun cas se faire au détriment de la protection des libertés

Qu'en est-il aujourd'hui ? Des expérimentations dont aucun bilan n'a été effectué sont désormais pérennisées, et à celles-ci s'ajoutent plusieurs nouvelles dispositions.

malheureusement, 58 des 59 attentats déjoués en France l'ont été par le biais du renseignement humain. La question de l'efficacité du renseignement automatisé demeure donc automatisé demeure donc pertinente. Le texte prévoit aussi l'extension des relations avec les opérateurs de communications électroniques, qu'il s'agisse de l'usage des à la faveur du déploiement de la 5G ou de l'interception des données satellitaires de proximité.

Comme à l'accoutumée pour ce type de texte très attentatoire aux libertés publiques, la commission des lois a toutefois joué son rôle de défenseur des libertés et droits fondamentaux en corrigeant le projet de loi pour anticiper les éventuelles censures constitutionnelles, s'agissant notamment des Micas, ou encore des mesures de rétention de sûreté. Je continue cependant de m'étonner de la persistance de la logique qui préside à cette inflation législative, celle-ci n'ayant pas fait les preuves de son efficacité. Mes chers collègues, les attentats terroristes de ces dernières années ont eu lieu sous le régime de ces mesures.

fragile. La complexité de cette question et la nature même des activités de renseignement appellent un débat de fond, à la hauteur de l'enjeu. Un tel

qui ont travaillé avec une diligence extrême sur un texte difficile, pour lequel le Parlement, singulièrement le Sénat, se trouve, si j'ose dire, « dans la seringue », par l'effet cumulé de décisions de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil d'État et d'une disposition votée à titre provisoire dont le délai de validité expire. Nous voilà donc contraints de décider de mesures multiples et importantes sans avoir eu le temps de les expertiser, et ce d'autant plus que le rapport sur les algorithmes, qui devait être remis au Parlement, le sera postérieurement à nos débats, ce qui, évidemment, ne contribuera pas Or ce texte est loin d'être anodin. Si l'on écoute nos collègues, en particulier notre excellent rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, tout est sous Il est vrai que les articles qui concernent l'utilisation des algorithmes- l'article 12 -, des drones- l'article 18 -, de la captation satellitaire et de la 5G sont indispensables à la lutte contre le terrorisme et à la protection de notre pays et de ses armées

pour les affaires qui ne seraient pas « graves » au sens de l'arrêt du Conseil d'État, mais qui peuvent être liées à la criminalité organisée ou aux trafics en tous genres, y compris d'êtres humains,

et la décision du Conseil d'État du 21 avril 2021, sans compter des recours pendants portant précisément sur l'article 15 à venir. Enfin, la question qui se pose et qui a été très justement relevée lors d'une table ronde organisée le 10 juin dernier par les commissions des lois et des affaires européennes du Sénat, est

De même, il faut rappeler qu'il n'existe pas de réglementation des activités des services secrets dans le droit de l'Union européenne, en dehors des questions relatives aux obligations de stockage et de transfert des données

pour des raisons de souveraineté, nous produisons ces algorithmes nous-mêmes et ne les achetons pas « sur étagère ». Pourriez-vous nous indiquer où en est le contrat avec Palantir,

plaidé pour une souveraineté numérique européenne face à la domination des États-Unis et de la Chine. Plus l'on donnera des moyens de contrôle à ces pays et moins l'on gardera de souveraineté. Et moins l'on aura de contrôle sur ces nouveaux outils de captation

impératifs qui brident le travail parlementaire et nous réduisent au rôle de chambre d'enregistrement. Il est extrêmement dommage que ce type de sujet

traite de la protection des Français face à la menace terroriste, du maintien de la compétitivité de nos services de renseignement au niveau international, du renforcement du contrôle parlementaire sur les services de renseignement et de l'accès aux documents d'archives classés secret-défense, afin notamment de favoriser le travail de recherche des archivistes et historiens. Je n'aborderai pas tous ces thèmes, laissant à ma collègue Chantal Deseyne le soin de s'exprimer sur le volet relatif au renseignement, en sa qualité de membre de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Je souhaite, pour ma part, mettre l'accent sur plusieurs dispositions introduites par les deux rapporteurs de la commission des lois, qui sont experts en la matière, Agnès Canayer, membre de la délégation parlementaire au renseignement, et Marc-Philippe Daubresse, qui assure depuis trois ans le suivi et l'évaluation de la loi du 30 Il s'agit donc du quatorzième texte en lien avec la sécurité et le terrorisme que le Parlement examine depuis les attentats qui ont sauvagement meurtri notre pays, en 2015 et en 2016. L'état d'urgence, instauré sur l'ensemble du territoire pour faire face à la menace terroriste élevée, a été prorogé à deux reprises.

Elle a permis l'expérimentation de quatre mesures exceptionnelles de police administrative dans le droit commun, afin de mieux prévenir les actes de terrorisme : les périmètres de protection, la fermeture de lieux de culte, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, ou Micas, les visites domiciliaires et les saisies. Ces mesures ont-elles montré leur efficacité ? Sans aucun doute. De plus, il est établi qu'elles ont fait l'objet d'une mise en oeuvre raisonnée et proportionnée. Ainsi, entre le 1 novembre 2017 et le 30 avril 2021, quelque 612 périmètres de protection ont été établis, 8 lieux de culte ont fait l'objet d'une fermeture administrative, 444 Micas ont été prononcées, 462 visites domiciliaires ont été réalisées, donnant lieu à 244 saisies. 57 visites domiciliaires ont fait l'objet de poursuites judiciaires, dont 30 pour des faits de terrorisme. Ces dispositions ont été prorogées en décembre 2020 pour sept mois, alors que la commission des lois du Sénat avait, à l'époque, proposé de les pérenniser, comme M. le rapporteur l'a rappelé. Aussi, nous Aussi, nous ne pouvons que souscrire à l'article 1, tout en regrettant amèrement que, une fois de plus, le Gouvernement et les députés n'aient pas accordé de crédit au travail du Sénat, retardant ainsi inutilement ces mesures tout à fait justifiées. Tout au long de l'examen du texte issu de l'Assemblée nationale, les rapporteurs ont veillé à assurer un équilibre entre les mesures de sécurité et le respect de l'État de droit et des libertés constitutionnelles. Ils ont également pris en compte les multiples réserves du Conseil constitutionnel sur plusieurs volets.

Or nous savons que 162 personnes condamnées pour actes de terrorisme devraient sortir de prison dans les quatre prochaines années. Il est donc nécessaire que puissent leur être imposées des mesures de surveillance et d'accompagnement à la réinsertion. En effet, comme le soulignait notre collègue Muriel Jourda, dans son rapport sur la proposition de loi de François-Noël Buffet renforçant le suivi des condamnés terroristes sortant de détention, les outils juridiques actuels ne sont pas satisfaisants. Ainsi, les rapporteurs ont introduit, à l'article 5, cette proposition de loi que nous avons votée en mai dernier et qui crée une mesure judiciaire de suivi et de surveillance. Celle-ci semble constituer une voie juridiquement plus adaptée que la proposition initiale du Gouvernement. En effet, cette mesure est prononcée par un juge, à l'issue d'une procédure contradictoire ; elle offre des possibilités de surveillance plus longues et plus contraignantes et permet d'associer aux obligations de surveillance des mesures sociales visant à favoriser la réinsertion de la personne. personne. Elle reprend le principe du dispositif adopté par le Parlement en juillet 2020, tout en y apportant les aménagements nécessaires pour répondre aux objections du Conseil constitutionnel. Par ailleurs, bien qu'ils approuvent différents ajustements du régime des Micas, les rapporteurs n'ont pas accepté l'allongement de leur durée à deux ans pour les personnes condamnées pour terrorisme sortant de détention.

Les rapporteurs ont également souhaité encadrer davantage le dispositif des périmètres de protection, en introduisant une autre réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, qui concerne la faculté pour les forces de l'ordre d'en contrôler l'accès, de procéder à des palpations de sécurité et de fouiller les bagages. Ils ont donc précisé que ces vérifications ne peuvent se fonder que sur des critères excluant toute discrimination, de quelque nature que ce soit, entre les personnes. Je terminerai par la question de l'accès aux informations relatives aux hospitalisations sans consentement des personnes inscrites au de la radicalisation à caractère terroriste, le FSPRT. Le Gouvernement prévoyait d'étendre de façon assez large la possibilité de communiquer ces informations aux représentants de l'État et à plusieurs services de renseignement. Les rapporteurs ont jugé que la diffusion de ces données devait être plus strictement encadrée et ont souhaité la limiter aux préfets et aux seuls agents placés sous leur autorité et spécialement désignés à cette fin. Madame la ministre, nous regrettons une nouvelle fois les délais contraints imposés au Parlement pour examiner ce texte très technique et complexe, en raison de la nécessité de l'adopter avant le 31 juillet 2021, date à laquelle les mesures de l'article 1 arriveront à expiration. Toutefois, je tiens à souligner la qualité du travail des rapporteurs, qui ont enrichi le texte tout en respectant l'équilibre entre mesures efficaces de lutte antiterroriste, respect des libertés fondamentales et conformité constitutionnelle. La commission des lois a suivi ses rapporteurs, ainsi que les rapporteurs pour avis, et elle a approuvé leurs propositions mesurées, efficaces et pragmatiques. Cependant, à la lecture des amendements déposés par le Gouvernement, je constate une fois encore que vous faites fi des apports du Sénat, en voulant rétablir en grande partie le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale. Qu'en est-il du respect du débat parlementaire si, dès la première lecture à la chambre haute, aucune discussion n'est possible ? L'enjeu de ce texte est majeur. Il faut renforcer notre arsenal législatif pour assurer la protection de nos concitoyens qui aspirent à vivre dans un État de droit, en toute sécurité. Ne l'oublions pas dans nos débats ! La parole est

Déjà, ils ont permis d'éviter de nombreux attentats sur notre sol. Ils vont parfois jusqu'à risquer leur vie pour protéger la nôtre : qu'ils soient ici remerciés de leur efficacité et de leur sang-froid. Nous en faisons le constat, depuis 2015, le terrorisme a évolué, passant d'une menace projetée des zones djihadistes à des agressions inspirées par la propagande, pour prendre désormais la forme d'une autonomisation totale de la menace, avec des acteurs isolés, au profil psychologique instable. Les causes et les risques ont changé, et les moyens d'efficacité ont évolué. Nous devons donc nous adapter. Nous y sommes Les évolutions technologiques permanentes entraîneront une nécessaire modification des contrôles. Ainsi, si l'utilisation des algorithmes se révèle encore plus indispensable qu'en 2015, il est nécessaire désormais d'utiliser les URL pour une plus grande efficacité. Sur ces sujets sensibles, la confiance est certes nécessaire, mais le contrôle démocratique l'est tout autant. Il arrive que nous soyons sur une ligne de crête entre liberté et sécurité, d'où la nécessité de considérer que la confiance n'exclut ni l'attention ni le contrôle.

Certes, dans cette hypothèse, le bicamérisme peut nous protéger, tout comme la délégation parlementaire au renseignement, la commission de vérification des fonds spéciaux, ou encore la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement,

car elles cherchent l'efficacité par l'adaptabilité. Nous devons cependant toujours être sourcilleux sur nos libertés fondamentales. C'est en ce sens que le Sénat et nous-mêmes jouons notre rôle, en faisant preuve d'attention À ce titre, je veux soumettre à votre sagacité deux sujets de vigilance, dont le premier concerne les échanges entre les services français et étrangers. Nous savons combien ceux-ci sont essentiels dans la lutte contre le terrorisme. Il serait néanmoins logique qu'il y ait un contrôle de ces échanges et que celui-ci soit exercé par une autorité indépendante, telle que la CNCTR. La plupart des pays européens le font, mais la France reste en retard. Les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme, le 25 mai dernier, devraient nous inciter fortement à revoir notre point de vue. En l'occurrence, il serait préférable d'anticiper une probable condamnation par la Cour européenne second point de vigilance porte sur la possibilité de voir le Conseil constitutionnel remettre en cause l'allongement des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, les Micas, ce qui, de plus, retarderait la mise en oeuvre rapide de la loi. Le Conseil d'État a émis des réserves. Il serait bon que le Gouvernement en tienne compte. Ce texte est nécessaire, comme son évolution le sera probablement aussi Notre assemblée et nous-mêmes souhaitons apporter des améliorations de précision et de précaution. Sur un tel sujet, le systématisme partisan n'est pas de mise.

ce projet de loi est pour notre pays d'une importance toute particulière. Il concerne, au premier rang, non seulement la sécurité des Français, mais aussi notre souveraineté. Le cyberespace a renouvelé en profondeur les modes d'action du renseignement. Cyberattaques, cyberespionnage, cyberguerres justifient une adaptation des règles de la sécurité nationale. La lutte contre le terrorisme demeure une priorité majeure. Les statistiques sur les techniques de renseignement relevant de la surveillance intérieure montrent que la prévention du terrorisme a motivé plus de 40 % des demandes soumises à l'examen de la CNCTR. La nécessité de répondre aux menaces et aux attentats terroristes a conduit le législateur à doter les services de renseignement de moyens d'investigation sophistiqués. La mise en oeuvre de ces techniques par les services de renseignement est définie de manière précise dans le code de la sécurité intérieure. Pour garantir sa légitimité, le renseignement doit non seulement convaincre de son efficacité, mais aussi déroger le moins possible aux valeurs démocratiques, ce qui suppose le respect de plusieurs principes fondamentaux, comme la séparation des pouvoirs, respect des règles de droit et la protection des libertés fondamentales. Ainsi, l'actuelle montée en puissance du renseignement doit s'accompagner du renforcement des contrôles qui pèsent sur la communauté du renseignement, au titre de l'indispensable exigence démocratique. Plusieurs évolutions législatives sont à l'oeuvre. L'article 6 étend la possibilité de communication des informations relatives à l'admission d'une personne en soins psychiatriques aux seuls préfets et agents placés sous leur responsabilité, lorsque celle-ci représente une menace grave pour la sécurité et l'ordre public, en raison de sa radicalisation à caractère terroriste. L'article 8 autorise la conservation des renseignements collectés jusqu'à cinq ans, à des fins de recherche et de développement, dans la perspective de permettre l'élaboration d'outils d'intelligence artificielle. Il prévoit la pérennisation de la technique de l'algorithme, qui permet l'identification précoce des menaces en se fondant sur l'analyse de l'ensemble de l'activité numérique de la population, pour repérer les comportements susceptibles de constituer un risque. Durant l'année écoulée, la CNCTR a constaté une augmentation des demandes d'accès aux données de connexion, conjuguée à une baisse des autres demandes, notamment celles qui sont relatives aux techniques les plus intrusives. Ce projet de loi prévoit d'intégrer aux données traitées par l'algorithme les noms de domaines consultés par les internautes. De la même façon, la surveillance en temps réel est étendue aux adresses complètes de ressources sur internet. La commission des lois du Sénat a considéré que cette extension ne saurait être inscrite de manière pérenne dans le droit, mais qu'elle pouvait être autorisée dans le cadre d'une expérimentation jusqu'au 31 juillet 2025. En raison du déploiement de nouvelles constellations satellitaires et du développement d'une offre étrangère de communication, l'article 11 autorise les services de renseignement, à titre expérimental, à intercepter par le biais d'un dispositif de captation de proximité les correspondances transitant par la voie satellitaire. Les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement sont renforcées. Les amendements adoptés par la commission des lois visent à prévoir que les recommandations et observations formulées par la délégation seront présentées au président de chaque assemblée. Les avancées proposées par ce texte sont nombreuses. Elles se justifient par le fait qu'il nous faut adapter le monde du renseignement aux évolutions technologiques dont se servent nos ennemis. Depuis la vague d'attentats de 2015, la menace d'une attaque projetée depuis l'étranger a laissé place à une menace plus diffuse, celle d'un terrorisme endogène. Jean-François Ricard, premier procureur du parquet national antiterroriste, expliquait lors d'une table ronde au Sénat que le travail effectué dans les enquêtes à caractère terroriste à partir des données de connexion représentait 80 % de l'activité des agents, dans le cas d'un attentat ou d'une association de malfaiteurs. Face à cette évolution, le rôle de la CNCTR est primordial. En 2020, la commission a rendu 262 avis défavorables, soit 0,8 % du nombre d'avis rendus. Je souhaite rappeler que, comme les années précédentes, le Premier ministre n'a accordé aucune autorisation après un avis défavorable de la commission. Parallèlement, ce projet de loi prévoit de renforcer le rôle de la CNCTR avec la mise en oeuvre de nouvelles dispositions. Ce texte est indispensable pour ceux qui, au sein des services secrets, travaillent à défendre les intérêts de la France et de ses ressortissants, partout où ils pourraient être menacés. Avant que nous ne commencions l'examen des articles, je tiens à rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui, dans le secret, travaillent à la protection des Français et de la République. La discussion La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la commission.

issues de la loi SILT, dont les rapports de contrôle parlementaire de l'Assemblée nationale et du Sénat ont présenté un bilan mitigé, mais bien à maintenir leur nature exceptionnelle. Nous tirons ainsi les leçons des mesures que le Sénat s'est lui-même appliqué à suivre et à préconiser dans le cadre de la crise sanitaire qui a bousculé nos libertés publiques. Au moment où nous sortons progressivement du régime de l'état d'urgence sanitaire contre l'épidémie de covid-19, l'honneur revient au Sénat d'avoir rappelé que la création de tout régime d'exception doit être limitée dans le temps, ce qui a conduit le Parlement à en fixer le terme au 31 décembre 2021. C'est l'une des leçons essentielles concernant les libertés publiques que le législateur devra retenir. En matière de législation d'exception, l'expérience montre qu'il existe une forme de paresse démocratique à introduire des dispositions dérogatoires au droit commun d'abord de manière expérimentale, pour les pérenniser ensuite, puis à en étendre le champ d'application au gré des circonstances. L'article 44 du projet de loi confortant les principes de la République, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, en témoigne de nouveau : il propose d'élargir le champ d'application de la fermeture des lieux de culte à partir d'autres fondements que le régime légal et provisoire d'exception et qui sont d'une gravité moindre. Pérenniser des mesures extrêmement dérogatoires au droit commun est un processus dont nous savons par avance qu'il conduit à rogner davantage le champ des libertés publiques. libertés publiques. Conscients de cette dérive, nous souhaitons maintenir le caractère exceptionnel des articles 1 à 4 de la loi du 30 octobre 2017. Ces mesures directement extraites du régime de l'état d'urgence accroissent de manière significative les pouvoirs de l'autorité administrative, avec pour seule finalité la lutte contre le terrorisme. pris en considération leur caractère expérimental, et à la suite des interventions ultérieures du législateur, qui a limité strictement leur champ d'application, le Conseil constitutionnel a jugé que ces mesures assuraient une conciliation qui n'était pas manifestement

Par ailleurs, dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, le Parlement a constaté que ces dispositions présentaient un intérêt en matière de prévention des actes de terrorisme et que, si leur appropriation par l'autorité de police administrative s'est révélée inadéquate à plusieurs reprises au moment de leur entrée en vigueur, leur utilisation actuelle semble mesurée et proportionnée. Il n'en demeure pas moins que ces mesures sont dérogatoires au droit commun, car elles affectent très clairement la liberté d'aller et venir, la liberté de culte, le droit au respect de la vie privée et familiale et l'inviolabilité du domicile, dans un contexte sécuritaire d'anticipation d'un danger potentiel. En conséquence,

les mesures de police administrative de la loi SILT de 2017. La commission des lois l'a adopté sans modification, puisqu'elle recommandait déjà dans ses travaux de pérenniser ces mesures, au moment où le Gouvernement avait décidé de les proroger, sous couvert de crise sanitaire, en décembre dernier. Je veux rappeler que le groupe CRCE s'était opposé à la loi SILT, qui est venue pérenniser un certain nombre de dispositifs issus de l'état d'urgence sécuritaire, déclenché à la suite des attentats de 2015. Cet article du projet de loi instaure donc définitivement la possibilité d'instaurer des périmètres de protection, les fermetures administratives de lieux de de culte et les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, les fameuses Micas. Ces dernières mesures administratives sont sans doute les plus graves. Elles peuvent être prononcées à l'encontre des personnes dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public, notamment.

infraction, mais sur la suspicion de la commission probable de cette infraction. Or les conséquences de ces dispositifs peuvent être très lourdes pour les personnes visées, qui sont jugées potentiellement dangereuses sur des critères extrêmement flous. Il s'agit là d'un tournant assez radical.

à l'Assemblée générale des Nations Unies, plusieurs États se sont inquiétés du manque de respect des droits humains dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en France. Ils ont insisté sur la nécessité de mettre en place un mécanisme

Il s'agit donc d'une déclinaison et d'un renforcement des mesures instituées en 2017. L'article prévoit ainsi la fermeture des locaux dépendant du lieu de culte fermé et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils seraient utilisés pour faire échec à l'exécution de cette mesure. Les motifs sont flous et viennent alimenter une police administrative de suspicion. En effet, le champ d'application très large de la mesure dépasse l'objectif de prévention et de lutte contre le terrorisme, et la notion de « locaux dépendant du lieu de culte » apparaît bien trop imprécise et susceptible de porter atteinte à la liberté du culte et à la liberté associative, d'autant plus si l'on considère que tous les dispositifs du projet de loi Séparatisme qui s'inscrivent exactement dans la même logique En outre, l'administration dispose déjà du pouvoir de dissoudre toute association incitant à la commission d'actes de terrorisme ou de fermer tout lieu constituant une menace pour l'ordre ou la sécurité publique. Pour toutes ces raisons, nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement de suppression. La

du code de la sécurité intérieure concernant les mesures de fermeture des lieux de culte. Cette disposition renforce les mesures d'une loi particulièrement délicate en matière de liberté d'exercice du culte, le but étant d'autoriser la fermeture des locaux dépendant du lieu de culte fermé dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils seraient utilisés pour faire échec à l'exécution de cette mesure. Il ressort de la rédaction de ce dispositif que le champ d'application de cette mesure est trop large, en ce qu'il dépasse l'objectif de prévention et de lutte contre le terrorisme, et que, par ailleurs, la notion de « locaux dépendant du lieu de culte » reste beaucoup trop floue. du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires estiment que cet article n'est pas compatible avec les principes de sécurité juridique et d'intelligibilité de la loi. Nous rappelons, en outre, que l'administration dispose déjà du pouvoir de dissoudre toute association incitant à la commission d'actes de terrorisme ou de fermer tout lieu constituant une menace pour l'ordre ou la sécurité publique. Dès lors, nous doutons de l'intérêt d'une telle mesure, qui paraît à la fois abusive et superfétatoire. Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de l'article 2, qui est susceptible de porter atteinte à la liberté du culte et à la liberté associative.

de la mesure de fermeture des lieux de culte, telle qu'elle est aujourd'hui prévue par l'article L. 227-1 du code de sécurité intérieure et telle qu'elle a d'ailleurs été validée par le juge constitutionnel. Les associations gestionnaires de culte disposent, dans la plupart des cas, de lieux dépendant du lieu de culte, que cette dépendance soit géographique ou qu'elle soit organique.

à l'origine de la fermeture initiale y soient diffusés, faisant ainsi échec à l'exécution concrète de la mesure de fermeture prévue. Par conséquent, il nous semble nécessaire de permettre la fermeture des locaux lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils seraient employés pour faire obstacle à la mesure de fermeture prononcée à titre principal. D'ailleurs, le Conseil d'État a reconnu, dans son avis sur le projet de loi, que cette disposition paraissait adaptée au but recherché, tout en satisfaisant les critères de nécessité et de proportionnalité, ce qui conserve intact l'équilibre entre la prévention des atteintes à l'ordre public

est ainsi libellé : La parole est à M. Ludovic Haye. Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l'article 2 dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale. En effet, la modification opérée en commission paraît procéder d'une vision à la fois trop large et trop restrictive de la notion de « locaux annexes au lieu de culte concerné Ainsi, le fait de viser tous les lieux gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne gestionnaire du lieu de culte dont la fermeture est prononcée conduirait à permettre la fermeture de locaux ne présentant aucun lien avec le motif de fermeture du lieu de culte. de culte. Cette portée du dispositif, sans lien avec la lutte contre le terrorisme, est, par nature, disproportionnée. À l'inverse, la mention « qui accueillent habituellement des réunions publiques » est, à nos yeux, un peu trop restrictive, car elle aurait pour effet d'exclure de nombreux locaux utilisés pour contourner la fermeture administrative, tels que les bibliothèques, les locaux associatifs destinés à l'accueil des enfants ou encore les centres culturels, qui n'accueillent pas habituellement de réunions publiques. Le rétablissement de l'article 2 dans sa rédaction initiale permettra d'empêcher les contournements d'une mesure de fermeture d'un lieu de culte, tout en garantissant la proportionnalité de la disposition. Quel

La mention des seuls « lieux accueillant des réunions publiques » nous paraît quant à elle trop restrictive, parce qu'elle exclut plusieurs lieux dépendant du lieu de culte dont la fermeture devrait pouvoir

et avec clause de rendez-vous, justement à cause de leur caractère particulièrement exorbitant du droit commun. Les Micas sont mises en oeuvre par le ministre de l'intérieur, après information du procureur de la République, à l'encontre de « toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ». Ces motifs sont particulièrement imprécis, difficiles à établir et à contrôler. s'agit en fait de la légalisation de ce que l'on appelle une « menace pressentie ». En effet, une personne faisant l'objet d'une Micas peut se voir imposer des restrictions importantes de liberté : assignation géographique et obligation de pointage auprès des services de police, interdiction de paraître dans certains lieux et signalement de tout déplacement à l'extérieur du périmètre défini. Dans les deux cas, le ministre de l'intérieur peut également prononcer une interdiction d'entrer en relation avec une ou plusieurs personnes. aujourd'hui, la durée des Micas est strictement encadrée, puisque celles-ci ne sont renouvelables que dans la limite d'une durée cumulée de douze mois et que, au-delà de six mois, des éléments nouveaux ou complémentaires sont requis pour les prolonger. Prétendant que, pour des profils présentant une dangerosité élevée, la limite de douze mois se révèle inadaptée, le Gouvernement souhaite, au travers de son amendement n° 89, rétablir le texte voté à l'Assemblée nationale, qui prévoyait un possible allongement à une durée de en précisant que, si le Conseil constitutionnel a fait de la limitation à douze mois l'un des éléments du bilan de la constitutionnalité de la Micas, il n'a pas été saisi de la différence objective de situation entre les personnes radicalisées n'ayant pas été condamnées et celles qui ont fait l'objet d'une condamnation. cependant, mes chers collègues, que le Conseil constitutionnel, dans le commentaire de cette même décision, a estimé que, quelle que soit la gravité de la menace qui la justifie, une telle mesure de police administrative ne peut se prolonger aussi longtemps que dure cette menace- c'était assez clair.

Monsieur le rapporteur, je prends acte de la position de la commission, qui refuse l'allongement du délai. Il n'empêche que l'article 3 pérennise les Micas.

L'amendement n° 89, présenté par le Gouvernement,

eux demeurent ancrés dans une idéologie radicale. Ces individus forment le haut du spectre des objectifs des services de renseignement et présentent des enjeux sécuritaires multiples à leur sortie de détention prosélytisme, menaces à court terme représentées par des profils impulsifs, menaces à moyen ou à long terme relatives à des projets d'attentats, tentatives de redéploiement vers les zones dites « de djihad » à l'étranger. L'expérience acquise au cours des dernières années nous permet aujourd'hui d'affirmer que le placement sous Micas constitue pour ces profils un outil particulièrement utile et adapté. Il permet de faciliter la surveillance d'individus qui sortent de prison, d'observer leurs relations habituelles volontaires, relations imposées qu'implique la détention, leur pratique religieuse, leur activité sur les réseaux sociaux, leurs efforts de réinsertion, etc., là où la mise en place d'une surveillance physique ou technique à temps plein se révélerait difficile, en raison notamment des ressources humaines qu'elle induirait.

depuis 2017 -, alors même que les services sont en mesure de justifier de la persistance de la menace constituée par le comportement des individus concernés. C'est la raison pour laquelle le projet du Gouvernement qui a été voté l'Assemblée nationale prévoyait, dans des conditions strictement encadrées, un allongement à une durée de deux ans. Votre commission des lois a souhaité supprimer cette possibilité, lui préférant un dispositif judiciaire qui reprend certaines obligations des Micas, comme l'interdiction de paraître ou l'interdiction de fréquenter certaines personnes. Cette solution ne semble pas convaincante à nos yeux, pour deux raisons principales. Premièrement, il nous semble que cette solution priverait les autorités de la réactivité nécessaire pour assurer le suivi des sortants de détention. L'expérience a en effet montré que les sorties de détention sont parfois décidées quelques heures seulement avant la sortie, ce qui ne place pas toujours l'autorité judiciaire en mesure de prononcer une mesure judiciaire, quand la Micas peut être prise par le ministre de l'intérieur en quelques heures seulement. Deuxièmement, la solution que vous proposez nous semble de nature à fragiliser fortement le recours à la Micas telle qu'elle est pratiquée actuellement et pourrait aboutir à une situation paradoxale, dans laquelle les personnes radicalisées qui ne seraient jamais passées à l'acte feraient l'objet d'un suivi plus strict que celles qui ont déjà été condamnées pour des faits de terrorisme. Pour ces raisons, le Gouvernement souhaite pouvoir rétablir la possibilité d'un allongement de la durée des Micas à vingt-quatre mois, telle qu'elle était proposée dans le projet de loi initial et qu'elle a été votée par l'Assemblée nationale. Je rappelle que cet allongement est encadré par des garanties fortes, qui permettent de sécuriser la mesure sur le plan

que les Micas, compte tenu de leur rigueur, ne sauraient, « sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, excéder, de manière continue ou non, une durée totale cumulée de douze mois le commentaire que le Conseil fait de cette décision, quelle que soit la gravité de la menace qui la justifie, une telle mesure de police administrative ne peut se prolonger aussi longtemps que dure cette menace.

alors que, comme je l'ai indiqué, les mesures judiciaires que nous proposons à l'article 5 présentent plusieurs avantages : elles sont prononcées par un juge, elles offrent des possibilités de surveillance plus longue et des garanties plus importantes pour les individus concernés et permettent d'associer aux mesures de surveillance des mesures sociales visant à favoriser la réinsertion.

mais je pense que la solution qu'il préconise ne nous permet pas d'en sortir et serait peut-être pire que le mal. La présence de témoins au cours d'une visite domiciliaire constitue une garantie essentielle du respect des droits de la défense et, d'ailleurs, du droit à un recours juridictionnel effectif. les témoins dans le procès-verbal, l'occupant des lieux ne disposerait plus d'aucun moyen de vérifier que ces témoins existent effectivement et que la visite domiciliaire a été effectuée dans le respect des prescriptions légales. M. Leconte propose

la présence de deux témoins lors de la visite domiciliaire en l'absence de la personne concernée est l'une des conditions de la régularité de la mesure. En effet, la copie du procès-verbal des visites domiciliaires et de saisie est transmise à l'occupant des lieux, pour que celui-ci puisse utilement, si d'aventure il le souhaite, exercer un recours. en l'absence de précisions sur l'identité des témoins qui auraient assisté à la visite domiciliaire, la personne n'est pas placée dans les conditions qui lui permettent d'apprécier la régularité de la mesure et, le cas échéant, de faire valoir ses droits. Pour ces raisons, l'anonymisation totale des témoins, sans aucune possibilité de voir leur identité révélée en cas de contestation, ne nous paraît pas possible. Le Gouvernement

Gréaume. Au travers de cet amendement, que nous avons souhaité insérer avant l'article 5 relatif aux mesures de sécurité, nous souhaitons engager la discussion sur les autres méthodes possibles en matière de lutte antiterroriste et de gestion des condamnés pour terrorisme. Pour ce faire, nous souhaitons que le Gouvernement remette au Parlement un rapport concernant les personnes détenues mises en cause dans des affaires de terrorisme islamique ou celles qui ont été écrouées pour des faits de droit commun et repérées par l'administration et les services de renseignement comme étant susceptibles de radicalisation. Ce rapport porterait sur les conséquences sur ces personnes de l'isolement et des quartiers spécifiques, de la réduction des aménagements de peine depuis la législation antiterroriste de 2016 et

Alors qu'ils étaient déjà rarement prononcés, la législation antiterroriste de 2016 est venue durcir les conditions d'octroi de certains de ces aménagements et en supprimer purement et simplement d'autres., c'est toute la philosophie de l'aménagement de peine, donc de la préparation à la sortie, qui est remise en cause. En outre, à partir de 2016, six quartiers d'évaluation de la radicalisation ont été mis en place sur tout le territoire. À la suite des évaluations menées, les personnes ancrées dans un processus de radicalisation violente et présentant une forte imprégnation idéologique et prosélyte sont affectées en quartier de prise en charge de la radicalisation, étanche du reste de la détention. Une telle situation concerne 15 % des détenus des quartiers d'évaluation de la radicalisation. Face à tout ce dispositif, dont les rouages semblent pourtant bien huilés, on nous propose aujourd'hui de déterminer un nouveau niveau de dangerosité et les mesures de sûreté appropriées, lorsque ces personnes ne seront plus écrouées.

pas de l'avis de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Aussi, plutôt que de faire de la surenchère sécuritaire pénale, il s'agirait peut-être de faire le point sur la méthode engagée pour lutter efficacement contre la récidive, en prenant le temps de réfléchir à la réinsertion de ces individus, plutôt qu'à leur exclusion. Quel

inévitablement conduit à l'existence de « sorties sèches », qui inquiètent tant, aujourd'hui, le Gouvernement, les parlementaires et, plus largement, la population dans son ensemble. Cet article tend à aménager le dispositif de régime de sûreté à l'encontre des détenus condamnés pour des actes de terrorisme et sortant de prison, voté l'été dernier et jugé non conforme à la Constitution dans la décision du Conseil constitutionnel du 10 août 2020.

Auparavant, le Conseil d'État s'était également interrogé sur l'utilité d'une telle mesure de sûreté. On peut ainsi lire, dans son avis du 23 juin 2020 : « La surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit permet l'application de presque toutes les mesures de la proposition de loi ». En effet, de nombreuses mesures de notre code pénal permettent d'ores et déjà d'assurer un suivi post-détention. On peut notamment citer le suivi socio-judiciaire prévu aux articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal, la mesure de surveillance judiciaire prévue aux articles 723-29 et suivants du code de procédure pénale, ou encore le suivi post-libération prévu à l'article 721-2 du code de procédure pénale. Si notre groupe prend très au sérieux la nécessité de prévenir la commission d'actes à caractère terroriste, la gravité de ces actes ne dispense pas d'apprécier la stricte nécessité des mesures prévues. Or, en l'état, la présente disposition, par ailleurs d'application rétroactive, je le je le souligne, porte une atteinte excessive aux libertés individuelles. C'est en tout cas l'avis du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, qui s'oppose à la mise en place de cette nouvelle mesure de sûreté. Nous regrettons également ne soit pas prise en compte la situation des prisonniers de droit commun qui se radicalisent au cours de leur détention. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression du présent article. Quel

tout à l'heure, l'amendement n° 87 a pour objet de rétablir la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion dans la version adoptée en première lecture. Afin d'assurer le suivi et la prise en charge de ces individus, le Gouvernement propose

réinsertion, afin de favoriser la réinsertion et de prévenir la récidive d'actes de terrorisme. Votre commission a jugé utile de réécrire intégralement l'article 5 du projet de loi, en créant une mesure judiciaire de sûreté mixte, qui comprend, d'une part, des obligations destinées à la réinsertion, comparables à celles qui étaient prévues dans le projet de loi du Gouvernement, des obligations destinées à assurer la surveillance de la personne, qui se rapprochent de celles qui étaient prévues par les Micas dans leur objet. Toutefois, le dispositif proposé par le Gouvernement

part, la surveillance de ces personnes, par le prononcé d'obligations et d'interdictions strictes, et, d'autre part, leur réinsertion, grâce à une prise en charge resserrée par des acteurs spécialisés de la réinsertion. Ce dispositif permet aussi une meilleure articulation avec les Micas, en évitant toute superposition des mesures administratives avec la mesure de sûreté judiciaire. Il conduit ainsi à renforcer la constitutionnalité de ces dispositions, qui doivent pouvoir être mises en oeuvre au plus vite. Je rappelle à cet égard que le Conseil d'État a constaté que le dispositif proposé répondait aux exigences posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 août 2020. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement souhaite le rétablissement de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste

n° 7 rectifié est retiré.

n° 22. L'article 6 autorise la communication aux préfets et à certains services de renseignements des données à caractère personnel issues du fichier relatif au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement, lorsqu'un patient représente une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics en raison de « sa radicalisation à caractère terroriste ». Le décret du 6 mai 2019 autorise déjà l'interconnexion de ce fichier OPCI web avec le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Une telle extension du nombre de personnes ayant accès à une information médicale contrevient aux principes du droit, au respect de la vie privée et au secret des informations médicales. Comme l'indique le Syndicat de la magistrature, la lutte antiterroriste, dotée d'un arsenal législatif pléthorique, continue à servir de prétexte à la création de toutes sortes de dispositifs exorbitants tels que le fichage et le traçage des personnes atteintes de troubles mentaux, sans qu'aucune corrélation ait été établie entre radicalisation à caractère terroriste et troubles psychiatriques. Dans la droite ligne des textes sur les responsabilités pénales et des mouvements de l'opinion publique sur le sujet, ce texte vient entériner l'idée que même les fous doivent être jugés,

présenter l'amendement n° 66. Le présent article tend à élargir au préfet et à certains services de renseignement l'accès aux informations relatives aux personnes admises en soins psychiatriques, et ce sans leur consentement. Rappelons tout de même que, à l'heure actuelle, seul le préfet de département est aujourd'hui autorisé à opérer une hospitalisation. Par Par cet élargissement, il s'agit d'assurer le suivi d'une personne représentant une menace grave pour la sécurité et l'ordre public. indiqué précédemment, nul ne peut dans cet hémicycle prétendre ne pas prendre au sérieux la menace terroriste. Il s'agit bien évidemment d'une cause nationale, qui requiert la mise en place de tous les moyens nécessaires à sa réussite, dans le respect des libertés fondamentales et dans la limite d'une atteinte injustifiée au droit des personnes. En l'occurrence, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires estime que la lutte antiterroriste ne doit pas servir de prétexte au fichage et au traçage des personnes atteintes de troubles psychiatriques. Tout d'abord, le secret médical a toute son importance et ne saurait être rogné par une énième loi sécuritaire. Ensuite, les phénomènes de radicalité violente sont compliqués et protéiformes. Nous affirmons donc fermement que ces dispositifs de contrôle stigmatisants n'ont pas leur place dans notre société.

Pour assurer leur suivi dans les meilleures conditions, il nous paraît nécessaire que les préfets des lieux de résidence, ainsi que les agents qui sont placés sous leur autorité, puissent avoir connaissance des entrées et des sorties. Le code de la santé publique permet d'ailleurs déjà aux préfets déjà aux préfets des départements d'hospitalisation de le faire. L'extension aux préfets des départements de résidence semble aller de soi. Pour autant, je connais l'argument,

défavorable à ces amendements, et ce pour une raison très simple. La commission des lois et la commission des affaires sociales ont fait un travail sur l'expertise psychiatrique et les difficultés

et de situation administrative de l'individu. Dans la mesure où le dispositif envisagé a pour objectif le seul suivi des personnes présentant une menace terroriste, ainsi que des troubles psychologiques ou psychiatriques, il nous semble indispensable que les services de renseignement puissent être destinataires de telles informations. Cela permet la prévention des passages à l'acte terroriste des personnes radicalisées présentant de tels troubles. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, dans lequel figure la question de la prévention du terrorisme. L'absence de communication aux services de renseignement pourrait conduire à nuire à cet objectif. Surtout, le dispositif de communication envisagé comporte plusieurs garanties. Tout d'abord, les finalités de cet échange d'informations sont limitées au seul sujet d'une personne qui présente une menace grave pour la sécurité et l'ordre public, à raison de sa radicalisation à caractère terroriste. Ensuite, outre le préfet, la communication se limite à une partie des services de renseignement services spécialisés ou « premier cercle », et seuls certains services du second cercle désignés par décret en Conseil d'État. Enfin, les échanges sont limités dans le temps, dans la mesure où les informations transmises ne peuvent porter sur des faits antérieurs de plus de trois ans à compter de la date de levée de la mesure de soins sans consentement. La parole

qui sont des services spécialisés, et des seuls services du second cercle, désignés par décret en Conseil d'État, aux informations sur les hospitalisations sans consentement. Il vise à présenter un certain nombre de garanties, qui viennent d'être développées par Mme la ministre, et le Conseil d'État n'a pas émis de réserves sur l'accès des services de renseignement à ces informations.

Pour montrer que nous sommes aussi soucieux d'efficacité, je serai favorable à l'amendement de repli de M. Haye et défavorable aux deux amendements identiques.

Le 9 septembre 1986, voilà maintenant trente ans, la France se dotait de sa première législation en matière de lutte antiterroriste. À l'époque, cette loi instituait un régime dérogatoire au droit commun, en créant un corps spécialisé de magistrats. Depuis lors, de nombreuses réformes ont conduit à la mise en oeuvre d'un régime procédural dérogatoire en matière d'enquêtes, ainsi qu'à la création de nouvelles infractions terroristes. À la suite des attentats du 13 novembre 2015, le conseil des ministres a adopté un décret déclarant l'état d'urgence. En à peine deux ans, cet état d'urgence a été prorogé six fois,

En juillet 2017, le président Macron nous promettait une unique loi sur le sujet, laquelle venait entériner des dispositifs issus directement de l'état d'urgence et de son régime exorbitant du droit commun. Cela se poursuit aujourd'hui avec cette nouvelle loi et ces nouveaux dispositifs. Ce texte va de nouveau très loin, comme l'ont souligné, dans une note d'alerte, les signataires du signataires du réseau Antiterrorisme, droits et libertés : « Le Gouvernement a perdu la boussole des principes de l'État de droit, en se réjouissant de l'hybridation des logiques administratives et judiciaires, et en considérant comme totalement superflu le principe selon lequel on ne saurait priver une personne de sa liberté

Le Parlement s'honorerait à mener ce travail à bien. Depuis 1986, les gouvernements successifs ont proposé des dizaines de textes dédiés à la lutte contre le terrorisme. Or jamais leur efficacité n'a été évaluée en termes de résultats. Ces dernières années ont été particulièrement marquées par le déploiement d'un arsenal pénal significatif : loi relative au renseignement, prorogation de l'état d'urgence, loi

De plus, dès lors qu'il intègre dans le droit commun des mesures qui suscitent l'inquiétude des associations de défense des libertés publiques, ce texte,

lutte le rapport budgétaire de politique transversale. L'orange budgétaire de politique transversale nous donne des évaluations, qui sont notamment liées au financement de l'ensemble des politiques de lutte antiterroriste.

La prévention des menaces communes auxquelles sont confrontés la France et ses alliés justifie pleinement la nécessité d'une coopération poussée entre les services de renseignement de ces différents pays. Il apparaît donc nécessaire de fixer un cadre à cette activité. un cadre à cette activité. La délégation parlementaire au renseignement avait estimé nécessaire en 2020 que cette réflexion soit lancée dans la perspective de l'examen du présent projet de loi, estimant qu'une réflexion était engagée dès lors que l'absence d'encadrement des échanges de renseignements étrangers pouvait constituer une source de fragilité juridique. Le Gouvernement s'était alors dit prêt à envisager un cadre réglementaire plus formalisé de ces échanges, notamment pour améliorer les conditions dans lesquelles les contacts avec les services partenaires étrangers sont établis.

l'avis de la commission ?

l'avis du Gouvernement ? de la Cour européenne des droits de l'homme relatives aux législations britannique et suédoise. Ces décisions appellent un examen minutieux pour mesurer leur implication sur la loi française, qui est très différente des lois de ces deux pays. La Cour se prononcera dans quelques mois sur notre législation. Il nous semble dès lors prématuré de tirer des conséquences dans notre droit de cette récente jurisprudence, qui ne concerne pas le droit français. Je souligne, au demeurant, que les dispositions de l'amendement n° 42 n'ont pas de portée normative. Il appartient en tout état de cause au Premier ministre, qui détermine et qui conduit la politique de la Nation, dispose de l'administration et est responsable de la défense nationale, de définir les orientations générales relatives à l'activité des services de renseignement et aux échanges avec leurs partenaires étrangers. l'amendement n° 43, quant à elles, posent une double difficulté. D'une part, cet amendement vise à supprimer la règle dite « du tiers service », garantissant qu'un renseignement reçu d'un service étranger n'est accessible à nul autre qu'à celui qui l'a reçu.

Or cela serait directement contraire à la séparation des pouvoirs, comme le rappelle d'ailleurs avec constance le Conseil constitutionnel. Je suis donc défavorable à ces deux amendements.

aujourd'hui des contrôles de ce qui se passe entre leurs propres services et les services étrangers. Les États-Unis, par exemple, ont une commission parlementaire spécifique du renseignement composée uniquement de parlementaires.

Attendre d'être allé dans le mur pour légiférer, ce n'est pas sérieux ! Il est absolument indispensable de commencer à le faire, même si c'est compliqué.

France est en retard sur les autres États occidentaux possédant des services de renseignement reconnus. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse, le Danemark, les Pays-Bas ou encore la Norvège sont dotés d'un contrôle spécifique, sans que cela nuise

d'informations à des partenaires de renseignement étrangers doit également être soumis à un contrôle indépendant », ce que son arrêt du 25 mai dernier a confirmé plus de trois ans après. Il apparaîtrait donc judicieux d'étendre les compétences de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui pourra ainsi vérifier le respect des orientations prises par le Premier ministre en la matière.

ministre. Ce sujet nécessite d'être travaillé en amont et réfléchi, eu égard aux conséquences, notamment sur le plan international et européen. Il importe également d'attendre les effets de la jurisprudence sur la législation française.

Mme Esther Benbassa. Le présent article acte la fin du principe selon lequel les renseignements ne peuvent être utilisés pour des finalités autres que celles qui motivent la procédure de surveillance. En effet, il prévoit la transmission de renseignements entre services et étend par là même la communication d'informations aux services de renseignement. Disons-le clairement, cet article est attentatoire aux libertés publiques. En permettant à des services de contourner les restrictions quant à l'usage de dispositifs de surveillance, la fin de ce principe de finalisation contrevient au droit au respect de la vie privée. De même, l'absence de contrôle préalable aux mesures de surveillance est problématique. 7 s'inscrit, de ce fait, dans la longue liste de dispositions poussant à la déjudiciarisation du contrôle en matière de sécurité intérieure. il interroge fortement quant à la traçabilité et à la durée de conservation de ces informations une fois transmises.

il n'est toujours pas sécurisé juridiquement, en l'absence de publication du décret d'application devant en préciser les modalités et conditions. En outre, il n'existe pas de dispositions particulières intéressant les renseignements pouvant être transmis au sein d'un même service.

de contrôle des techniques de renseignement ne soit pas un avis conforme. Au regard des techniques utilisées, particulièrement intrusives, il est essentiel qu'une autorité indépendante donne un avis contraignant. La Commission nationale Renforcer le contrôle de la CNCTR, afin de le rendre effectif, est primordial pour qu'elle dépasse son rôle de faire-valoir des décisions de l'exécutif. Compte tenu du caractère extrêmement attentatoire aux libertés et à la vie privée des pouvoirs qui seraient donnés aux services, des garanties doivent être prévues, afin de protéger les libertés individuelles de nos concitoyens. C'est pourquoi le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires souhaite rendre l'avis de la CNCTR conforme. Mme Esther Benbassa. Les interceptions de masse réalisées par les services secrets danois sur les communications électroniques transitant par ce pays montrent qu'il est urgent

rendu public le 25 mai dernier, la Cour européenne des droits de l'homme précise les conditions dans lesquelles les interceptions de masse réalisées par les services secrets sont acceptables à ses yeux. À l'aune de cet arrêt, une condition majeure n'est pas remplie par la France en raison de l'absence totale de contrôle, qu'il soit politique ou juridique, de l'échange de données avec les services de renseignement étrangers. Un tel vide législatif interroge. Qui contrôle la conformité au droit des échanges entre la communauté française du renseignement et ses partenaires étrangers Qui s'assure que sont respectées les libertés individuelles de nos concitoyens ? Ni le Parlement ni l'autorité judiciaire ou,, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement n'ont de droit de regard sur ces sujets.

Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise donc à combler un angle mort de la réglementation encadrant les services de renseignement. Quel

est un article d'équilibre. Il vise à encadrer un certain nombre d'échanges, notamment pour les renseignements utilisés avec une finalité différente de celle pour laquelle ils ont été autorisés, ainsi que la transmission de renseignements à des services qui n'auraient pu y avoir accès

d'autant que celui-ci sera également examiné dans les prochains mois par la Cour ; nous ne savons pas, au préalable, ce qu'elle en dira. Au demeurant, nous considérons que vous donnez une portée excessive à l'arrêt. Pour ce qui est de la transmission de renseignements à un service étranger partenaire, la Cour de Strasbourg n'impose nullement une autorisation préalable par une autorité indépendante. Nous ne sommes donc pas d'accord avec les fondements mêmes de cet amendement. Par conséquent, l'avis du Gouvernement

l'avis de la commission ?

sont détruites dès lors qu'elles ne sont pas ou plus nécessaires à l'accomplissement des missions du service auquel elles ont été transmises ». Cette disposition ne nous semblant pas assez précise, nous proposons d'ajouter les mots : « et au plus tard dans un délai de six mois ». En effet, nous considérons que les services de renseignement ne doivent

M. Yannick Vaugrenard. L'examen de ce projet de loi était l'occasion de traduire en droit la réflexion promise sur l'encadrement juridique des échanges entre les services de renseignement français et ceux de nos partenaires étrangers. Nous considérons qu'il s'agit en quelque sorte de l'angle mort du projet de loi et avons déposé des amendements visant à remédier à cette situation, en proposant un encadrement de ces échanges sous la tutelle du Premier ministre

Démocratie et Territoires, vise à élargir les compétences de la CNIL à l'ensemble des fichiers échappant à son contrôle. Il existe aujourd'hui treize fichiers ayant trait à la sûreté nationale sur lesquels aucun contrôle n'est exercé par la CNIL. La préservation d'un strict équilibre entre la sécurité publique, la protection des intérêts fondamentaux de la Nation et le respect de la vie privée nécessite des garanties et le contrôle d'une autorité indépendante du pouvoir politique.

enjoignent d'apporter une garantie supplémentaire à nos concitoyens, afin que les protections de la loi Informatique et libertés soient pleinement appliquées. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires demande une modalité de contrôle renforcée de la CNIL.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Je voudrais ajouter que ces fichiers de souveraineté n'échappent pas au droit. Ils font l'objet de formalités préalables à leur création, qui permettent à la CNIL et au Conseil d'État de se prononcer sur la conformité des conditions de leur mise en oeuvre. En pratique, l'avis que la CNIL donne sur le projet de texte autorisant le traitement lui permet aussi d'apprécier les caractéristiques du fichier et leur conformité à la loi Informatique et libertés. La CNIL s'assure ainsi, en particulier, que les catégories de données collectées, la désignation des accédants et des destinataires de ces données, ainsi que les éventuelles interconnexions, soient adéquates, nécessaires et proportionnées aux finalités du fichier. Enfin, il est inexact de prétendre que la mise en oeuvre de ces fichiers, une fois autorisée dans les conditions que j'ai rappelées, échapperait à tout contrôle. Les modalités de collecte des données conservées dans ces fichiers de souveraineté font l'objet d'un contrôle dédié au titre de la mise en oeuvre de techniques de renseignement, sous l'égide de la CNCTR. La CNIL est très régulièrement amenée, par des contrôles ciblés effectués sur ces fichiers au sein même des locaux des services de renseignement, à s'assurer de l'existence, de la pertinence et de la proportionnalité des données concernant toute personne qui l'a saisie à cette fin au titre du droit d'accès indirect. Ce contrôle permet d'ailleurs d'obtenir, le cas échéant, l'effacement des données qui auraient été irrégulièrement collectées. Je rappelle que nous avons eu, voilà quelques mois, le débat sur la question des « fichiers liberté » ici même, au Sénat. pour ces fichiers de souveraineté permet de concilier les impératifs liés à la sûreté de l'État et les droits des personnes concernées. Introduire un pouvoir de contrôle général, de surcroît, de la CNIL sur ces fichiers n'est donc ni souhaitable, ni efficace, ni nécessaire

l'avis de la commission ?

déjà de manière exhaustive les intérêts fondamentaux de la Nation, parmi lesquels figure, bien évidemment, la prévention du terrorisme. Même si elle n'est pas explicitement mentionnée, la lutte contre ce fléau dans toutes ses composantes est concernée,